d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, alors que la République se bat pour maintenir son autorité sur l'ensemble du territoire national, alors que nos forces de l'ordre font face à une dangereuse montée en puissance de la délinquance et de la violence, et alors que nos concitoyens subissent quotidiennement les effets de l'insécurité, la Défenseure des droits a une idée pour le moins saugrenue : expérimenter des zones sans contrôle d'identité. Cette proposition est ahurissante : pourquoi ne pas exploiter des zones sans policiers, des zones sans pompiers, et, finalement, des zones sans droit ? Ce dont souffrent notre pays et nos concitoyens, c'est non pas d'un trop grand respect de la loi mais de son insuffisante application. Notre pays et nos concitoyens souffrent du désordre, du manque de respect de certains pour la loi et l'autorité. Mme la Défenseure des droits a le droit de défendre le droit, et bien sûr le droit des gens à vivre en sécurité. Dans leur immense majorité, les Français sont bien conscients de la nécessité de lutter contre cette insécurité qui les menace. Ils savent que les forces de l'ordre interviennent avec beaucoup de difficultés dans certains quartiers, et ils ne demandent pas moins de police, bien au contraire. La discrimination n'a pas sa place dans notre pays, dans notre République. Mais la proposition de Mme la Défenseure des droits n'est qu'un renoncement, une République à deux vitesses où les lois s'appliqueraient selon les quartiers. Elle contient une insinuation insupportable : elle laisse entendre qu'un contrôle d'identité se ferait forcément au faciès et qu'il faudrait arrêter ces contrôles. Policiers et gendarmes remplissent leur mission avec exemplarité, et ceux qui manquent à leurs devoirs sont sévèrement punis. Nous voulons assurer ici aux forces de l'ordre tout notre soutien. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que cette expérimentation n'aura pas lieu, car il est vital d'assurer l'autorité de l'État dans tous les territoires de la République.

comme vous le savez toutes et tous, la Défenseure des droits, autorité pour laquelle nous avons beaucoup de respect, est une autorité administrative indépendante (AAI) qui formule un certain nombre de préconisations. Il se trouve que le Gouvernement de la République est également indépendant de la Défenseure des droits ! Très bien ! Avec tout le respect dû, je le répète, à cette institution, je dis solennellement devant le Sénat et devant le pays qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de zones sans contrôle d'identité, en application des lois de la République. La parole

En effet, les murs des facultés ne sont pas extensibles, pas plus que les terrains de stage ou le nombre des enseignants chargés de former Néanmoins, la loi de 2019 promettait de mettre fin au gâchis des abandons après redoublement ; elle promettait de diversifier le parcours des recrutements

Il semble en effet qu'un flou persiste sur le nombre de places réellement ouvertes et que, dans certaines facultés, le nombre de places déjà réservées aux redoublants de la Paces

Là encore, la plus grande place a été donnée aux discussions entre les universités, les ARS et les acteurs locaux pour définir le nombre de places offertes en deuxième année d'études de santé ; ce nombre a évidemment été augmenté par rapport à l'année dernière, puisque c'est une obligation. Comment les choses se mettent-elles en place ? Pour les redoublants de la Paces ancienne version, il nous est apparu important de maintenir un nombre de places équivalent, en moyenne, à la réussite des trois dernières années des redoublants dans

La ville de Trappes est à la une des médias. Pour avoir été maire de la ville voisine et président de la communauté d'agglomération dont Trappes fait partie, je suis meurtri par la stigmatisation médiatique dont cette ville fait l'objet. rénovation urbaine (ANRU), des centaines de millions d'euros ont été investis, des immeubles démolis puis reconstruits, tandis que des équipements publics sont flambant neufs. Le changement visuel est évident, mais hélas, les problématiques sont toujours là et s'intensifient dans certains quartiers ... Une véritable pandémie, avec un variant islamiste particulièrement nocif. Toutefois, il ne faut pas résumer Trappes à cela, car un véritable travail est fait sur le terrain entre les représentants de l'État et les élus locaux. Nous ne voudrions pas voir ces efforts anéantis par les déclarations tonitruantes d'un professeur, d'un maire qui tente de défendre sa ville, certes, mais qui se permet de distribuer des documents dans l'enceinte d'un lycée, de personnes menacées de mort qui sont aujourd'hui sous protection policière et de partis populistes qui surfent sur la vague en cette période préélectorale. Cette polémique éclate alors que l'on ne compte plus les flambées de violence un peu partout sur le territoire : à Besançon, avec une agression raciste ultraviolente ; à Montbéliard, avec des actes de sauvagerie et de guérilla urbaine sur lesquels ma collègue Annick Jacquemet souhaitait aussi vous interpeller à Paris, avec le lynchage abominable du jeune Yuriy ; à Poissy, avec un guet-apens couplé à un appel au meurtre, pour ne citer que les plus récents. Face à ces situations, la police semble dépassée.

Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le Premier ministre, que le Gouvernement va réagir avec les moyens nécessaires au climat d'incivilité qui sévit dans certains quartiers, partout en France ? La parole est à M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le

il n'est pas question pour le Gouvernement de désigner un territoire plutôt qu'un autre. Étant moi-même l'élu d'un territoire difficile, je sais combien les élus, les acteurs associatifs et les enseignants, combien tous ceux qui concourent à donner toute sa beauté à une ville, même lorsqu'elle est confrontée à des problèmes, voient parfois leurs efforts ruinés par un événement médiatique.

les policiers, dès le lendemain de l'agression, sont retournés sur le terrain et ont pu interpeller deux personnes. Oui, les territoires de la République sont parfois attaqués et, bien évidemment, nous devons renforcer les moyens matériels et humains de la police. Nous devons surtout redire que l'autorité est au coeur du pacte républicain et qu'elle doit chaque fois l'emporter, à Trappes comme ailleurs.

Dans cet hémicycle, nous sommes nombreux à participer à des collectes alimentaires pour leur apporter, dans l'extrême urgence, des moyens de subsistance dont beaucoup sont cruellement privés. Avant la pandémie, près de la moitié des étudiants travaillaient pour pouvoir étudier. Aujourd'hui, la très grande majorité d'entre eux est privée de ces emplois. Votre gouvernement vient d'annoncer la prolongation de la prime versée aux salariés intermittents, qui n'ont pu travailler correctement en 2020 160 000 jeunes de moins de 30 ans qui vont bénéficier de cette mesure. Le Président de la République a déclaré qu'un étudiant devait avoir les mêmes droits qu'un salarié. Pourquoi les étudiants ont-ils été exclus de ce dispositif ? Votre gouvernement vient d'annoncer le versement d'une prime de 1 000 euros pour aider les jeunes à payer leur loyer. Les jeunes apprentis en alternance pourront bénéficier de cette prime. bénéficier de cette prime. Pourquoi les étudiants ont-ils été exclus de ce dispositif ? Monsieur le Premier ministre, pourquoi la politique du « quoi qu'il en coûte » s'est-elle arrêtée systématiquement à la porte des campus ? porte des campus ? La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Peut-être pourriez-vous demander au CNRS de lancer une enquête sur ce sujet Madame la ministre, 40 % des étudiants qui pouvaient retourner à l'université ne l'ont pas fait, et vous considérez que c'est parce qu'ils préfèrent l'enseignement à distance. Je crains qu'ils n'y reviennent jamais ! Pour éviter ce désastre, c'est maintenant que le Gouvernement doit agir

L'économie sociale et solidaire (ESS), c'est aujourd'hui 10 % de notre PIB et 2,4 millions de salariés. Pour la seule région des Hauts-de-France, dont je suis issu, cela représente 180 000 emplois salariés et plus de 11 800 établissements employeurs. Toutes ces Toutes ces entreprises ont un grand potentiel d'innovation, car elles sont ancrées dans le territoire et sont de parfaites réponses aux besoins ou aux opportunités. Qu'il s'agisse de l'urgence sanitaire, alimentaire, éducative ou tout simplement citoyenne, des solutions innovantes ont, depuis plusieurs mois, été trouvées par toutes les coopératives et entreprises sociales dans notre pays, en coopération avec les autorités locales. Oui, la crise actuelle souligne autant le rôle nécessaire des acteurs de la solidarité aujourd'hui, que le besoin de transformer le modèle économique en s'inspirant des pratiques et des valeurs de l'ESS demain. Dans l'après-covid, il sera nécessaire de promouvoir la coopération en offrant les services de base d'une manière différente, en rétablissant et en créant des emplois décents grâce à des modèles d'organisation de la production divers et complémentaires.

Il y a urgence à sauver ce secteur, notamment toutes ces petites structures que nous connaissons bien sur nos territoires, qui font assaut d'imagination et de volontarisme dans leurs actions quotidiennes, mais qui, pour nombre d'entre elles, ont bien du mal à maîtriser les arcanes des dispositifs déployés par le Gouvernement. L'urgence est là, madame la secrétaire d'État, et je sais que vous y êtes particulièrement sensible. À l'aune de cette crise sans précédent, ma question sera donc simple : quelles mesures ont été mises en place pour sauver le soldat ESS ? La

c'est le non-recours aux aides qui sont à disposition de ces structures de l'ESS. C'est pourquoi, en plus de leur indiquer ce à quoi elles ont droit, je m'attelle à leur expliquer comment

Monsieur le secrétaire d'État, comme vous le savez, en plein milieu de la pandémie, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a été victime, la semaine dernière, d'une cyberattaque massive de son système informatique, alors même que celui-ci était conforme aux exigences réglementaires du programme HOP'EN. De telles attaques sont désormais trop banales. À Dax, les médecins n'avaient plus accès à l'historique des dossiers des patients. Les calculs de dose pour la chimiothérapie n'étaient plus possibles. Il a fallu faire ces calculs à la main, ce qui a limité la capacité de traitement quotidienne. Même si le fonctionnement a été sous-optimal, j'ai été impressionné lors de ma visite par l'engagement sans faille de l'ensemble des agents, un engagement qu'il faut saluer. Toutes les équipes se sont mobilisées, conscientes de l'urgence d'assurer le maintien du service public. C'est ce qui a permis de réduire les pertes de chances pour les patients. La professionnalisation de ces attaques comme des attaquants est un fait incontestable. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) signale une augmentation de 255 % de ce type d'attaque en 2020. Le secteur de la santé est particulièrement touché. Le CHU de Bordeaux subit ainsi une vingtaine de cyberattaques chaque jour. Cette cybercriminalité est à la hauteur de ce qu'elle peut rapporter : les demandes de rançon varient entre 200 000 et 10 millions de dollars. En parallèle, les coûts en matériels et en personnels dédiés sont de plus en plus importants, pour les structures privées comme publiques. Cette situation rapidement décrite m'amène, monsieur le Localement d'abord, si l'ARS et l'Anssi ont tout de suite été au chevet de l'hôpital de Dax, celui-ci mettra du temps à récupérer. Pouvez-vous me garantir son accompagnement vers un retour à la normale, y compris s'agissant des répercussions financières engendrées par l'attaque ?

d'État, voilà bientôt un an que nous vivons avec le virus et les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie. Cette situation a modifié en profondeur les habitudes de nos concitoyens et n'a pas épargné le secteur du loisir, qu'il soit sportif ou culturel. De multiples activités étaient auparavant proposées partout en France, parfois par des entreprises privées, mais le plus souvent par les communes ou par des associations. Chacun ici connaît et reconnaît le formidable travail de ces bénévoles associatifs, trop peu nombreux, portant souvent à bout de bras leur structure, sacrifiant leurs loisirs et leur vie de famille. Avec la fermeture au public des lieux de pratique, les adhérents se sont tournés vers d'autres activités plus individuelles, y compris vers des supports informatiques ou numériques. Certains ont demandé le remboursement des cotisations, mettant les associations en difficulté financière. De nombreux dirigeants associatifs, à bout de souffle, pensent abandonner. Des animateurs, désemparés et inquiets, s'interrogent sur leur avenir. Demain, la fanfare ou la reprendront-elles après des mois d'inactivité ? L'école de musique ou le club de théâtre vont-ils redémarrer ? L'association sportive retrouvera-t-elle ses adhérents ? Les moyens financiers seront-ils suffisants pour poursuivre ? Autant de questions qui inquiètent dans nos villages comme dans nos quartiers urbains. Toutes ces activités sont le ciment de notre société. Elles créent du lien social et du vivre ensemble. Au moment où le Parlement débat du séparatisme, nous sommes plus que jamais conscients de leur nécessité. Madame la secrétaire d'État, je souhaite savoir si vous partagez ces inquiétudes et connaître les mesures que vous envisagez pour permettre à ces structures, toutes différentes, mais toutes nécessaires, de ne pas disparaître.

à la biomasse de la tranche 4 de la centrale à charbon de Provence, située sur les communes de Meyreuil et de Gardanne. Depuis l'annonce de la fermeture de la tranche 5 charbon d'ici à 2022, l'État tente de mettre en place un pacte de territoire pour l'avenir du site industriel, qui inclurait la méga-centrale et des projets classés Seveso en plein coeur d'une zone urbanisée. Depuis 2017, après l'accord conclu entre l'État et Uniper, l'industriel repreneur s'est engagé à fournir 7 500 heures d'électricité par an, que l'État rachètera trois fois le prix du marché. Un tel procédé ne pourrait-il pas s'apparenter à une subvention déguisée de 1 milliard d'euros pendant la durée du contrat ? Ce site rencontre des difficultés techniques pour fonctionner, au-delà des mouvements de grève connus par le passé. L'industriel ne remplit toujours pas ses obligations en matière de fourniture de

est à Mme la ministre de la transition écologique. Monsieur le sénateur Benarroche, comme vous le signalez, le Président de la République s'est engagé à fermer les dernières centrales à charbon d'ici à 2022. C'est un pas important sur le plan écologique : nous économiserons ainsi l'équivalent des rejets de CO2 de 4 millions de véhicules. Bien sûr, la fermeture des centrales implique de donner aux territoires concernés de nouvelles perspectives de développement. Nous le faisons, main dans la main, avec les collectivités, les partenaires sociaux et les associations, à travers les pactes territoriaux. Vous citez la centrale de Gardanne. Vous n'ignorez pas que cette décision de politique énergétique, que vous soutenez, n'est pas aisée à mettre en oeuvre. Disons-le : des emplois sont supprimés sur le site de la centrale, comme auprès des sous-traitants et sur le grand port de Marseille-Fos. C'est une difficulté supplémentaire sur le territoire de Gardanne. C'est pourquoi nous avons apporté des solutions complémentaires, à travers des crédits supplémentaires de l'État et un accompagnement social renforcé des salariés. Enfin, nous n'avons pas souhaité ajouter de la difficulté aux difficultés. En effet, la centrale de Gardanne-Meyreuil compte une tranche biomasse, autorisée il y a près de dix ans maintenant, par le gouvernement de l'époque. Le contrat de rachat de l'énergie produite suit un mécanisme classique, correspondant à l'ancienne politique de soutien à l'électricité produite à partir de biomasse. J'y insiste, ce n'est pas une spécificité de Gardanne : plusieurs dizaines de lauréats ont été désignés entre 2005 et 2019, à l'issue d'appels d'offres. Certes, le contrat de rachat prévoit des pénalités si l'installation n'atteint pas une disponibilité minimale ; mais, dans le cas de Gardanne, il a été jugé que la longueur, l'ampleur et les causes de la grève qui a paralysé le site ces dernières années justifiaient de ne pas les appliquer pour les années 2018 à 2020, ce qui explique la situation que vous mentionnez

De plus, cette centrale se trouve dans un bassin industriel à l'avenir obscur, avec les boues rouges aux incidences écologiques préoccupantes- toujours acceptées par votre gouvernement -, et au devenir économique incertain après le rachat de l'usine par une entreprise guinéenne. J'attendais aujourd'hui une position du Gouvernement sur l'aspect concurrentiel ou non de cette méga-centrale biomasse et des précisions sur un contrat qui reste opaque. Enfin, j'aurais aimé apprendre du Gouvernement la véritable nature des relations liant sa politique énergétique au propriétaire, le groupe EPH du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, acquéreur de nombreuses centrales à charbon en Europe, ... Il faut conclure. ... intéressé par l'énergie lorsqu'elle est subventionnée par l'État et par ailleurs repreneur de nombreux médias français

Protéger, c'est aussi respecter la dignité humaine des personnes âgées et vulnérables. Cette dignité dans la vie ne peut pas être bafouée au motif de sauver des vies. Protéger, c'est aussi gérer la fin de vie. Nous devons permettre à la famille d'accompagner son parent jusqu'au bout. Protéger, c'est lutter contre le virus de la solitude. Le fait de vieillir enfermé entraîne un véritable risque de glissement pouvant conduire jusqu'à la mort, avec le refus brutal de communiquer, de s'alimenter et de recevoir des soins, malgré le dévouement exemplaire des personnels. Monsieur le ministre, le tout-sanitaire n'a-t-il pas atteint sa limite aujourd'hui ? Quelles perspectives et quelles solutions proposez-vous pour rompre avec cette situation mortifère ?

je vous remercie de votre question, qui me permet d'aborder un sujet éminemment humain, au-delà des enjeux sanitaires. Face à un virus qui nous était inconnu- vous en conviendrez -et qui frappait notamment les personnes âgées

La réalité, malheureusement, est que la France fait partie des pays les moins avancés dans la vaccination. Plutôt que d'autosatisfaction, faites preuve d'humilité et d'efficacité

La crise sanitaire et économique a encore accentué les inégalités, la précarité et les difficultés financières des plus modestes. Or, pour beaucoup de nos concitoyens, cette situation sociale est aggravée par les pratiques des établissements bancaires, qui continuent, l'air de rien, de prélever chaque mois leurs commissions diverses, frais de gestion et frais pour incidents de paiement. Après une légère baisse ces deux dernières années, le montant moyen des frais bancaires est de nouveau à la hausse.

La mécanique des frais bancaires est une mécanique appauvrissante dont il est difficile, voire impossible, de s'extraire. Ces frais représenteraient une manne financière

Aujourd'hui, alors que la pauvreté explose dans notre pays, l'urgence sociale exige que vous n'attendiez plus pour protéger les Français de frais bancaires opaques, excessifs et injustes. Ma question est donc simple : allez-vous enfin agir pour mettre fin à ces abus ?

un plafonnement à 25 euros par mois de tous les frais d'incidents pour les clients fragiles. S'y ajoute un plafonnement à 20 euros par mois et à 200 euros par an des frais d'incidents pour les bénéficiaires de l'offre spécifique clientèle fragile, que les banques doivent proposer à leurs clients en situation de fragilité. Nous avons aussi obtenu des banques qu'elles s'engagent à accroître de 30 % le nombre de bénéficiaires de cette offre spécifique, et cet engagement est tenu : l'augmentation a même

pour les publics à faibles revenus, qui connaîtraient des incidents répétés, ou en situation de surendettement. Enfin, nous avons exigé des établissements bancaires la pleine transparence quant à leur appréciation des publics fragiles. Depuis mai 2020, la Banque de France a mis en place une cellule d'alerte en cas de difficultés rencontrées par un particulier en matière d'inclusion bancaire et d'application de frais bancaires. Ainsi, depuis 2017, le Gouvernement, avec le concours des parlementaires, a fait davantage pour réduire réduire les frais d'incidents bancaires appliqués aux publics fragiles qu'aucun gouvernement auparavant. Plus que des engagements, nous pouvons invoquer des résultats. En un mot, en 2019, 1,4 million de Français avaient déjà vu leurs frais bancaires totaux réduits ! Tout cela

les Français les plus modestes s'appauvrissent et les frais bancaires augmentent. Je vous le répète : agissez et reprenez notre proposition de loi, adoptée par le Sénat

Mme Claire Hédon, ancienne journaliste nommée Défenseure des droits il y a peu par le Président de la République, imagine suspendre les contrôles d'identité dans certaines zones en France, car elle juge ceux-ci « insupportables pour certains jeunes ». Ainsi, pour Mme Hédon, l'État ne pouvant pas lutter efficacement contre la délinquance dans certains secteurs de notre pays, il vaudrait mieux démissionner, mettre son coeur en bandoulière et créer un cadre juridique spécifique afin d'assurer la pleine sérénité de ceux que la justice, la police et la gendarmerie irritent et dérangent. Pourquoi ne pas créer des « fan zones » réservées aux délinquants et entièrement sanctuarisées pour que les honnêtes gens n'y entrent surtout pas ? la violente attaque des forces de l'ordre par une bande de jeunes à Poissy, au cri de « Tuez-les ! », a certainement fait vaciller les certitudes de Mme Hédon. Ainsi, face au tollé provoqué par sa proposition, la Défenseure des droits est revenue hier sur ses dires, tout en réaffirmant cependant qu'il existe des « contrôles d'identité discriminatoires Cette position est surréaliste. Elle incarne le penser faux et le renoncement qui gangrènent la France depuis de trop nombreuses années. années. Monsieur le Premier ministre, vous venez de clarifier la position du Gouvernement. Mais, au-delà de cette actualité, pensez-vous réellement que le rôle du Défenseur des droits soit de jeter l'opprobre, de lancer des anathèmes sur nos forces de l'ordre, déjà suffisamment attaquées et éprouvées ces derniers temps

nous avons d'ailleurs constaté qu'elle les avait quelque peu corrigés -et il est évident que le ministère de l'intérieur ne mettra pas en place une telle expérimentation. Il est évident que les contrôles d'identité sont nécessaires.

le travail de la police que de le souligner. C'est mal connaître le travail des forces de l'ordre que de ne pas voir que les contrôles d'identité sont toujours menés sous l'autorité, soit du procureur de la République et donc du pouvoir judiciaire, soit d'un officier de police judiciaire, soit de policiers, lorsqu'ils constatent qu'un crime ou un délit Faisons confiance à nos forces de l'ordre. C'est le cas des parlementaires, représentants de la Nation ; c'est le cas du ministre de l'intérieur, vous le savez ; c'est le cas du Gouvernement tout entier ; c'est le cas du Président de la République et c'est le cas de l'immense majorité des Français.

Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé des transports. Elle porte sur l'articulation entre défense de l'environnement et développement des grandes infrastructures, en partant de l'exemple du contournement est de Rouen. En septembre 2017, après quasiment cinquante ans d'études, la région Normandie, le département de la Seine-Maritime, que je présidais à l'époque, et la métropole Rouen Normandie ont conclu un accord pour boucler le financement du contournement est de l'agglomération rouennaise. est indispensable. Rouen est la seule métropole française de cette taille- plus de 500 000 habitants -à ne pas bénéficier aujourd'hui d'une telle infrastructure. Or, le 8 février dernier, le nouveau président de la métropole a décidé d'y renoncer sous la pression de ses alliés écologistes. C'est un véritable électrochoc. La région et le département ont donc pris l'engagement d'accroître leur participation financière pour couvrir le renoncement de la métropole. L'État est le maître d'ouvrage de cette infrastructure. Jusqu'à présent, la réalisation du projet était soumise à la participation de toutes les collectivités concernées. L'État va-t-il y renoncer parce que la métropole s'en est retirée ou bien va-t-il mener à son terme un engagement que le Conseil d'orientation des infrastructures (COI) et la loi d'orientation des mobilités (LOM) ont identifié parmi les plus importants pour le développement de notre pays ? Plus globalement, l'exemple rouennais pose la question de l'articulation entre infrastructures et protection de la nature. On ne peut pas opposer les premières à la seconde par principe. En l'occurrence, un contournement fluide entraîne moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un engorgement urbain permanent- parle même pas de l'aspect sanitaire du problème, car la qualité de l'air s'en ressent pour les habitants. L'inscription de la protection de la biodiversité dans la Constitution

à l'époque -, le département de la Seine-Maritime et la région de Normandie, avaient quant à elles confirmé leur engagement financier en 2017, pour 50 % de la subvention d'équilibre, et l'État devait prendre en charge l'autre moitié du financement. Ces dispositions étaient effectivement inscrites dans la LOM. Néanmoins, comme vous le mentionnez, d'importants débats se sont élevés lors des élections municipales de 2020 à Rouen, au regard des enjeux généraux de protection de l'environnement et des besoins des habitants, qu'il s'agit évidemment de concilier : nous sommes tous d'accord sur ce point. M. le préfet de région avait alors demandé aux collectivités de confirmer leurs intentions. Le département et la région ont renouvelé leur soutien quand la métropole a fait part de son désengagement financier de l'opération et proposé d'autres solutions. Nous avons bien pris note du souhait de la région et du département de prendre en charge les 66 millions d'euros initialement dévolus à la métropole. Nous suivons ce dossier avec une attention particulière, mais

au dialogue entre les parties prenantes. Nous sommes prêts à étudier sérieusement toutes les propositions qui sont soumises pour concilier ces deux nécessités absolues : d'une part, la mobilité des habitants de la métropole et des personnes qui la traversent, de l'autre, la protection de l'environnement.

Depuis maintenant huit ans, nos forces armées sont déployées au Sahel. Le courage, l'abnégation et la compétence de nos soldats ont permis d'y remporter de nombreux succès militaires et d'empêcher la constitution d'un sanctuaire islamiste. Les défis à relever restent cependant considérables. Face à un ennemi toujours dangereux et en perpétuelle mutation, nos armées devront en permanence adapter leur dispositif opérationnel, mais aussi pouvoir s'appuyer sur la montée en puissance des forces armées de nos partenaires pour contrer efficacement la menace. Face à un ennemi qui se nourrit des fragilités et des défaillances des États de la région, la paix et la sécurité ne pourront renaître à la seule faveur d'une action militaire. Les conditions de cette renaissance sont par ailleurs économiques et politiques. Ce n'est qu'en progressant sur cette voie que l'on pourra durablement consolider les acquis de l'opération et conjurer la tentation d'un retrait précipité, qui ruinerait tous les efforts et les sacrifices consentis.

que le sommet de N'Djamena devait être celui « du sursaut diplomatique, du sursaut politique et du sursaut du développement ». Ces trois volets sont en effet indispensables pour redonner des perspectives, et d'une certaine manière du sens, à l'engagement de nos troupes sur le terrain. Monsieur le secrétaire d'État, quels ont été, lors de ce sommet, les messages adressés par le Président de la République à nos partenaires ? Estimez-vous qu'ils ont permis de provoquer ces sursauts que vous appelez de vos voeux ? La parole

Le Président de la République a participé au sommet du G5 Sahel, ou sommet de N'Djamena, par visioconférence, au début de cette semaine, lundi et mardi. Il a également pris

Vous l'avez souligné : il était temps de faire le point sur ces engagements et d'amplifier la dynamique amorcée. Le Président de la République a eu l'occasion de le dire publiquement : le sommet de N'Djamena a permis de dresser ce bilan, d'enregistrer des résultats et des réussites dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, il a indiqué un certain nombre d'avancées très concrètes,

Compte tenu de cet alignement politique et militaire, et de l'implication accrue de nos partenaires africains et européens, le Président de la République a indiqué que nous maintiendrions notre effort militaire et que, si des évolutions devaient être apportées, nous les examinerions en temps voulu, après l'amplification de cette dynamique.

La parole est à Mme Claudine Lepage, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Un peu partout sur le territoire, l'inquiétude, voire la colère, des enseignants et des parents d'élèves du second degré gronde. En cause, les discussions autour de la dotation horaire globale, qui doit acter votre choix budgétaire de supprimer 1 800 emplois d'enseignants dans le second degré. Ce choix conduit de nombreux établissements à préparer la rentrée scolaire dans des conditions intenables. Alors que votre gouvernement proclame à longueur d'interviews la priorité donnée à la jeunesse, cette mesure va emporter des conséquences désastreuses sur la qualité des enseignements : classes surchargées, restriction des choix d'enseignements, recours trop important aux heures supplémentaires, réduction du nombre de professeurs remplaçants, etc. Notre jeunesse, durement touchée par les conséquences de l'épidémie de la covid-19, sera la victime collatérale de ces suppressions de postes incompréhensibles. Incompréhensibles, car la situation sanitaire devrait, au contraire, nous conduire à recruter davantage d'enseignants pour diminuer le nombre d'élèves par classes et mieux les encadrer. Incompréhensibles, car la réforme du lycée que vous avez souhaitée nécessite des moyens en heures et en postes. Monsieur le ministre, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vous avait déjà alerté sur les conséquences que vos choix budgétaires allaient emporter sur le terrain, mais il n'est pas trop tard pour agir pour agir ! Allez-vous entendre la colère des enseignants et des parents d'élèves, revenir sur votre décision et prévoir, à l'inverse, des mesures exceptionnelles d'accompagnement pour la rentrée 2021 ?

le meilleur taux d'encadrement à l'école primaire. C'est le résultat d'un choix politique très fort : la priorité donnée à l'école primaire. Disons-le très clairement, la France dépensait jusqu'à maintenant moins que la moyenne des pays de l'OCDE pour son enseignement primaire et davantage pour son enseignement secondaire.

le devenir du canal du Midi, qui proposait des modifications de l'organisation et de la stratégie afin de préparer la réhabilitation et d'assurer la vie de ce grand site historique, patrimonial, paysager et très fortement touristique pour notre grande région.

fortement. Votre ministère a en effet réduit de façon drastique, depuis plusieurs années, les crédits dédiés au fonctionnement général,

région Occitanie et pour la France, pour leur attractivité historique. Par ma réponse, je voudrais simplement vous rassurer, si vous étiez inquiet, quant à l'implication très forte de l'État aux côtés des collectivités territoriales, non seulement pour la sauvegarde, mais aussi pour la restauration

et 75 millions d'euros sont prévus globalement dans le plan de relance. Pour ce qui concerne les investissements, j'ai signé avec la présidente de la région Occitanie il y a quelques semaines, à Tarbes, un accord de relance extrêmement ambitieux qui, s'agissant de l'État

territorial auquel le Gouvernement et votre serviteur sont particulièrement attachés. Oui, le canal du Midi a un avenir ; oui, il contribuera au développement économique, écologique et touristique de la région Occitanie

en novembre dernier, avec mes collègues du Grand Est, nous vous faisions part de notre vive préoccupation quant à la situation de Strasbourg, siège du Parlement européen. Nous appelions à des actions fortes du Gouvernement pour défendre et conforter la place de la capitale française de l'Union européenne. Cela fait désormais un an qu'aucune session plénière du Parlement européen ne s'est tenue à Strasbourg, et nous venons d'apprendre que la session de mars ne s'y tiendrait toujours pas ! C'est une atteinte aux traités européens et au principe de l'Europe polycentrique, au coeur même de l'idée européenne. La tenue des sessions plénières à Strasbourg ne saurait être optionnelle et la pandémie, qui concerne aussi bien la Belgique que la France, ne saurait plus longtemps être un prétexte pour remettre en cause la vocation européenne de Strasbourg. Actuellement, le format hybride des sessions plénières est piloté non depuis Strasbourg, mais depuis Bruxelles, avec près de 350 à 450 députés présents physiquement à Bruxelles. Le Parlement européen a tenu vendredi dernier, depuis Strasbourg, un exercice de simulation parlementaire rassemblant plus de 2 500 jeunes, preuve qu'il est parfaitement capable de piloter en ligne un événement qui dépasse le nombre de députés européens participant aux sessions plénières. Fin janvier, le Conseil de l'Europe a tenu, en présence physique et à distance, son Assemblée parlementaire avec des élus venus de quarante-sept États membres, dans de parfaites conditions d'organisation. Ce qui est possible pour le Conseil de l'Europe doit l'être pour le Parlement européen. Monsieur le Premier ministre, vous nous aviez indiqué votre total engagement pour défendre la vocation européenne de Strasbourg, mais les paroles ne suffisent plus. Nous ne pouvons plus assister passivement à cette situation et nous limiter à des réactions à chaque remise en cause du statut de Strasbourg. Face à une situation qui ne saurait perdurer, pouvez-vous nous dire ce que compte faire votre gouvernement pour permettre aux députés européens de revenir enfin dans la capitale européenne ? La parole

partage, au nom du Gouvernement et sous l'autorité du Premier ministre, votre préoccupation et vous assure de notre total engagement, rappelé par le Président de la République lui-même, pour un retour le plus rapide possible des sessions du des sessions du Parlement européen à leur siège prévu par les traités, qui se situe à Strasbourg. Cela n'a que trop duré. La situation sanitaire pose d'évidentes difficultés, mais elle ne saurait justifier ce type de comportements et la situation qui perdurera jusqu'à la session du mois de mars. Nous poursuivrons les démarches diplomatiques au plus haut niveau auprès du président du Parlement européen, M. David Sassoli, le Premier ministre en avait pris l'engagement en répondant au courrier que vous aviez porté avec un certain nombre d'autres élus. Je relaierai de nouveau ces messages lors des prochains jours. Vous savez que la situation du Parlement européen est

partagé que nous consacrons au statut de Strasbourg, nous sommes en train de finaliser entre l'État et les collectivités territoriales un nouveau contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne », qui verra les moyens financiers ceux de l'État- nous en avons pris l'engagement -mais aussi, nous l'espérons, ceux des collectivités territoriales impliquées. Je tiendrai une nouvelle réunion dans les prochains jours avec l'ensemble des élus de tous bords

de capitale européenne. Vous savez également qu'un hommage sera rendu au Parlement européen au président Valéry Giscard d'Estaing dans les prochaines semaines. Ce sera l'occasion de réaffirmer cette vocation européenne le plus solennellement possible. Nous

cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des finances a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable (13 voix pour, 1 voix contre) au renouvellement de M. Patrick de Cambourg à la présidence de l'Autorité des normes comptables. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de deux missions d'information : l'une relative aux conditions de la vie étudiante en France ; l'autre intitulée : « La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts. » Conformément à l'article 8 de notre règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques ont été publiées. Elles seront ratifiées s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par le règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

C'est un fait. Signées le 13 juillet dernier à Matignon, ces revalorisations profitent à l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux de l'hôpital, notamment public. Au-delà de ces revalorisations, attendues depuis bien longtemps par-delà les âges et les alternances, le Ségur de la santé a permis de dresser un diagnostic solide et partagé de l'ensemble de notre système de santé. Nous n'avons éludé aucun sujet : investissements, pour regarder l'avenir avec confiance ; gouvernance, pour redonner le pouvoir à ceux qui soignent- en tout cas, partager les processus de décision

Après l'Assemblée nationale voilà quelques semaines, le Ségur de la santé franchit donc à nouveau les portes du Parlement. S'il était indispensable de donner la parole aux soignants, il ne l'était pas moins que les représentants de la Nation s'emparent d'un sujet qui concerne tous nos concitoyens. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour le travail d'enrichissement et de consolidation que vous avez mené en commission et qui, je n'en doute pas, sera poursuivi dans cet hémicycle.

Cette proposition de loi répond également à la revendication, ancienne et renforcée par la crise sanitaire, visant à laisser une plus grande liberté d'organisation interne des établissements de santé à la main des acteurs locaux. La crise a montré que les collectifs de soins savaient s'adapter, s'organiser et surmonter des situations extrêmement sensibles sans attendre un accord, une validation ou un feu vert venu d'en haut.

Nous devons continuer à progresser en matière de démocratie hospitalière. À cet égard, ce texte prévoit de faire siéger au sein du directoire des établissements publics hospitaliers un représentant des personnels non médicaux, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers.

Certains membres de la commission des affaires sociales se sont inquiétés, émus même, du manque d'ambition de ce texte, notamment en matière de gouvernance, craignant des dissonances normatives et une forme d'insécurité juridique. Je tiens à rassurer chacun

de commission médicale de groupement (PCMG) sont revues dans l'ordonnance, ainsi que certaines recommandations du rapport Claris, qui ont fixé le cap que nous suivons. La réforme de la gouvernance hospitalière, j'y tiens ; elle est en train de se dessiner, avec celles et ceux qui, demain, présideront aux destinées de l'hôpital public dans notre pays.

la situation peut devenir proprement scandaleuse. Pour qui connaît la vie d'un service, c'est aussi et surtout une plaie qui mine la cohésion de toute une équipe. Par ailleurs, ce texte renforce un certain nombre de mouvements nés l'été dernier, avec le Ségur de la santé.

c'est faire le choix de la confiance et de l'efficacité ; c'est faire le pari que notre système de santé ne relèvera pas les défis qui l'attendent en ménageant les guerres de chapelles et les prés carrés.

nous devons trouver ensemble les voies et moyens par lesquels les mesures décidées l'été dernier trouveront à s'appliquer concrètement, sur le terrain, dans les territoires, dans chaque service hospitalier de France.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, faire confiance et simplifier : l'intitulé de cette proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, est riche de promesses. La crise sanitaire a contribué, depuis un an, à inscrire ces objectifs fédérateurs au coeur des attentes des acteurs de santé. Exprimée tant dans le Ségur de la santé que dans la mission sur la gouvernance hospitalière présidée par le professeur Claris, leur aspiration, légitime, est de se recentrer sur leur coeur de métier : le soin. le choc de confiance et de simplification tant attendu n'est clairement pas au rendez-vous de ce texte. La commission en a déploré le contenu disparate et, sur certains volets, chétif, le prisme et le manque de vision stratégique. cette proposition de loi ne nous paraît pas porter haut l'ambition pour notre système de santé que ses acteurs de première ligne, au front de l'épidémie depuis un an, sont aujourd'hui en droit d'attendre. Cette ambition appellerait, selon moi, la discussion d'un texte à l'ossature plus forte, plutôt que procédant à des ajustements. Surtout, la cohérence de certaines mesures que nous sommes appelés à examiner est mise à mal par le calendrier

aux contours indéfinis : engagée, je crois, sans concertation avec les professionnels intéressés, cette mesure n'avait pas sa place dans un texte censé rétablir la confiance avec les acteurs.

des associations dans l'encadrement des bénévoles qui interviennent dans le contexte, si sensible, des lieux de soins, en refusant les dérives que pourrait entraîner la notion de bénévole individuel. concerne les dispositions relatives à la gouvernance hospitalière, je ne puis vous cacher, monsieur le ministre, que la déception de la commission est réelle.

soient, pour la plupart, des traductions, parfois édulcorées, des recommandations émises par le professeur Claris au terme de sa mission sur la gouvernance hospitalière ou issues de la concertation du Ségur de la santé. La possibilité de former une commission médico-soignante, le droit d'option en matière d'organisation interne, la recomposition du directoire, le plan de gouvernance et de management et même la lutte contre l'intérim médical sont autant de mesures dont l'annonce produit certes un effet de courte durée,

avons supprimé l'article 4 , le considérant comme une véritable provocation à l'égard des praticiens hospitaliers, dont la vie privée subissait une atteinte manifestement disproportionnée. a fait part de son intérêt pour plusieurs initiatives qui seront discutées en séance en ce qui concerne l'inégalité de traitement entre l'activité libérale exercée par un praticien hospitalier d'un établissement public de santé

Elle a sécurisé les compétences du chef de service afin d'éviter tout chevauchement avec celles des chefs de pôle. Elle a fait droit à la demande très ancienne d'approfondir la délégation de gestion au sein de l'établissement. Enfin, elle s'est attelée à traiter l'une des causes du défaut d'attractivité de l'hôpital public pour les personnels paramédicaux. Mes auditions ont montré qu'il est en grande partie lié à un défaut de représentation auprès de la direction. avons donc prévu l'inscription de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) au rang des organes représentatifs de l'établissement public de santé, ainsi que l'élection de son président par ses membres.

de tous bords politiques, servant la construction d'un hôpital public moins contraint et plus soucieux d'assurer à ses personnels l'attractivité qui lui fait aujourd'hui tant défaut.

au problème, désormais structurel, de l'abandon résigné de l'hôpital public par nos gouvernements successifs, la commission a une nouvelle fois rappelé qu'aucune mesure législative ne pourrait durablement se substituer aux revalorisations salariales qui s'imposent. L'urgence est là, impérieuse. Mais avec le mauvais génie français de la réforme, il semble que les évidences les plus criantes restent encore ignorées

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe a fait le choix de déposer cette motion tendant à opposer la question préalable, car nous sommes opposés aux orientations de cette proposition de loi. D'ailleurs, soignants comme non-soignants sont vent debout contre la plupart des mesures qu'elle contient. Monsieur le ministre, vous avez utilisé la proposition de loi de la députée Stéphanie Rist pour compléter certaines mesures du Ségur de la santé, L'adoption de ce texte serait lourde de conséquences pour notre système de santé- des conséquences bien éloignées de la volonté de simplification affichée ... Ainsi, il s'agit notamment de renforcer l'échelon des groupements hospitaliers de territoire, qui devient davantage encore la référence, alors même que le rapport de la Cour des comptes d'octobre dernier est plutôt mitigé. proposition de loi offre une place prépondérante aux gestionnaires et technocrates, ceux-là mêmes qui ont conduit l'hôpital public à l'asphyxie. Parallèlement, ou paradoxalement, le texte autorise le bénévolat à l'hôpital, ce que mon collègue député Pierre Dharréville a comparé, à juste titre, à une forme d'ubérisation des activités associatives. Notre groupe a déposé cette motion car nous nous opposons au texte non seulement sur le fond,

Cette méthode présente l'avantage pour lui de l'exonérer d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État, ce qui laisse de fortes incertitudes sur les conséquences de ce texte que nous refusons. Le plus grave est le décalage entre ce texte et le vécu des professionnels de santé et du médico-social. Comment oublier que ce texte, présenté comme le prolongement du Ségur de la santé, fait suite à la première vague de covid-19 et, surtout, à des mois de mobilisation de collectifs et de syndicats des personnels ?

Alors qu'il faudrait s'attaquer aux racines du malaise des personnels soignants- manque de moyens, pilotage comptable, gestion calquée sur le privé -, ce texte prolonge une vision libérale de l'hôpital public en assumant l'introduction des règles du management privé dans le secteur public.

au mépris de l'histoire du service public hospitalier, des valeurs incarnées par ses agents et des services rendus aux populations dans le respect de l'égalité de toutes et tous, quels que soient l'origine sociale et le territoire. Derrière l'argument des contraintes organisationnelles se dissimulent l'autonomie de gestion et l'autonomie de moyens des établissements de santé. L'autonomie n'est donc qu'un paravent pour justifier, pour justifier, plus tard, une baisse supplémentaire des dépenses de l'État ou de la sécurité sociale. De plus, en renforçant l'autonomie des hôpitaux, vous forcez la main aux réorganisations des services et des métiers administratifs et techniques. Il faut au contraire renforcer l'égalité d'accès aux soins, plutôt que de casser le cadre national du service public de santé en prenant modèle sur l'autonomie des universités, qui a aggravé la mise en concurrence des établissements et encouragé le financement privé. La crise semble ainsi vous fournir un prétexte pour aller plus loin dans la déréglementation. Vous ne le faites pas au hasard : vous le faites pour pousser le plus loin possible les logiques gestionnaires et technocratiques qui ont contribué à affaiblir l'hôpital public. Voilà qui va encore alimenter la mise en concurrence des structures et favoriser la gestion pyramidale et centralisée des hôpitaux.

Alors que les bilans financiers démontrent l'échec des groupements hospitaliers de territoire, vous décidez d'accélérer ce que vous appelez l'intégration par l'installation de méga-GHT. Pourtant, les personnels que je rencontre lors de mes nombreux déplacements dans les hôpitaux et les Ehpad publics l'ont toujours fait, de remettre en cause ce pilotage à distance par des superstructures. Redonner de l'attractivité aux professions de la santé et du médico-social passe par la revalorisation des métiers et l'augmentation salariale, mais aussi par le partage des pouvoirs et donc des décisions. la réhabilitation des chefs de service est totalement amoindrie par le maintien des pôles. Pourquoi ce maintien, alors que la majorité des professionnels, à l'image du collectif interhôpitaux, demandent leur suppression, critiquant la bureaucratie qu'ils engendrent ? ? , ce que vous appelez la gouvernance doit redonner à chacune et à chacun sa place et s'appuyer sur deux piliers : la fin des politiques d'austérité, avec un objectif national des dépenses d'assurance maladie à la hauteur,, de de l'évolution naturelle des dépenses ; et l'instauration d'une véritable démocratie sanitaire, avec une représentation plus importante de l'ensemble des professionnels médicaux, administratifs et techniques, des étudiantes et étudiants internes de médecine, des usagers et des élus locaux, totalement absents des prises de décision.

donc une offre de soins égale pour l'ensemble des territoires. Ainsi, les centres de santé sont totalement oubliés. Pourtant d'après les chiffres du Conseil national de l'ordre des médecins, le nombre de médecins exerçant au moins une partie de leur activité en centre de santé

notamment chez les généralistes. Il est donc nécessaire de renforcer l'attractivité des centres de santé, qui assurent l'accès aux soins non programmés que les médecins libéraux ont abandonnés depuis le décret Mattei supprimant les gardes les nuits, les week-ends et les jours fériés.

Mme Buzyn y avait répondu par la suppression du dans les études de santé. Mais sans moyens supplémentaires accordés aux universités, sans investissements immobiliers et sans revalorisation du tutorat, cela revient à la situation actuelle de stagnation du nombre de médecins formés. Selon Emmanuel Vigneron, géographe de la santé, plus on est loin, moins on a d'informations et moins il y a de médecins. Pourtant, la crise sanitaire de la covid-19 souligne l'enjeu que constitue l'investissement dans l'éducation à la santé et dans un maillage territorial d'accès aux soins. malgré deux éléments positifs- la suppression de l'article 1, qui créait des professions médicales intermédiaires, article vilipendé de tous ; le maintien de plusieurs articles renforçant les prérogatives des sages-femmes et contribuant ainsi à une meilleure reconnaissance de cette profession médicale

Le plus grave, monsieur le ministre, est qu'aucun enseignement n'a été tiré de la pandémie que nous vivons depuis près d'un an et qui ne s'éteint toujours pas. Vous continuez à prendre des mesures dans le droit-fil des réformes qui ont conduit notre système de santé là où il en est aujourd'hui- loi HPST de Roselyne Bachelot, loi Santé de Marisol Touraine, loi Ma santé 2022 d'Agnès Buzyn -, avec en supplément la casse du cadre national du service public de santé.

s'explique par la faible prise en compte des enseignements issus des rapports de la Cour des comptes et du professeur Claris et, surtout, de la mobilisation qui s'est produite, pendant la pandémie, autour des longues négociations du Ségur de la santé. Il s'agit donc pour le Gouvernement de passer en force en prenant le risque d'avoir simulé la concertation, consentie il est vrai sous la pression de la mobilisation des professionnels de santé, pour poursuivre selon la même logique : celle qui fragilise encore et toujours notre système de santé et affaiblit l'hôpital public, lequel, en pleine pandémie, perd encore des lits.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, certaines manières de légiférer installées par l'actuelle majorité gouvernementale étaient déjà très contestables avant l'irruption de la covid-19 dans nos vies. La crise sanitaire les rend encore plus difficilement supportables, quand il s'agit de réformer dans la précipitation le système de santé, comme c'est le cas avec la présente proposition de loi. de loi. Très insatisfaisante sur le fond, celle-ci atteste la constance du mépris exprimé par l'exécutif aussi bien à l'encontre du Parlement que des partenaires sociaux. Tels sont les constats qui motivent la motion demandant le renvoi à la commission que je présente aujourd'hui au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat. Il y a en effet beaucoup à redire quant au traitement réservé au Parlement et au travail législatif. La genèse, le contenu et les modalités d'examen de la présente proposition de loi

La proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification est censée traduire dans notre droit les mesures non budgétaires annoncées dans le cadre du Ségur de la santé. Il aurait été opportun que ces mesures fassent l'objet d'un projet de loi et non d'un texte d'origine parlementaire. Il s'agit pour l'exécutif d'obtenir la transposition dans la loi d'un certain nombre des dispositions du Ségur de la santé, mais en se soustrayant aux contraintes qui sont liées à l'élaboration et à l'examen d'un texte d'origine gouvernementale. En procédant de la sorte, le Gouvernement se libère de deux obligations : le texte n'a fait l'objet ni d'un avis du Conseil d'État ni d'une étude d'impact. Pourtant, le respect que nous devons aux soignants aurait exigé qu'un tel texte soit non seulement sécurisé juridiquement par un avis du Conseil d'État, mais qu'il fasse également l'objet d'une étude d'impact afin que ces conséquences soient analysées. Les études d'impact ne sont décidément pas le fort de ce gouvernement : on se souvient de celle qui accompagnait le projet de loi portant réforme des retraites, étrillé par le Conseil d'État. Cette proposition de loi se veut pourtant ambitieuse. Par conséquent, elle est susceptible d'affecter lourdement un système de santé dont nous avons plus que jamais besoin qu'il fonctionne efficacement. Je m'interroge donc sur le sens des circonstances et l'appréhension par la majorité de la gravité de ses responsabilités et de ses obligations. Elle improvise sans méthode et sans rigueur la réforme d'un système de santé dont le bon fonctionnement est aujourd'hui plus que jamais impératif. C'est pourtant le moment de bien faire les choses ou de ne pas les faire. Nous n'y sommes pas Les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estiment que les dispositions que porte cette proposition de loi ne sont pas inscrites dans le bon véhicule législatif. Celui-ci pose d'emblée problème

Ce n'est pas un hasard si la majorité des professions concernées par cette proposition de loi sont vent debout contre ses dispositions, qui ont également suscité la profonde indignation des syndicats et des professionnels de santé, et un rejet unanime de la part de l'ensemble des acteurs.

relatif à la création d'une profession médicale intermédiaire, puis à sa suppression pure et simple dès le stade de l'examen en commission au Sénat. Ce manque de concertation relève d'une méthode et traduit une conception très descendante de la politique. Elle joue des tours au Gouvernement, car elle se manifeste notamment par un recours accru aux ordonnances et aux mesures réglementaires qui empiètent excessivement sur le domaine du Parlement. Ainsi, la commission des affaires sociales n'a pas manqué de souligner le paradoxe consistant pour le Gouvernement à promouvoir des dispositions qui ont aussi fait l'objet d'ordonnances et de mesures réglementaires. Les dispositions déjà modifiées par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, promulguée il n'y a même pas deux mois et demi, le sont, par ailleurs, de nouveau dans cette proposition de loi. Il en va de même pour les dispositions concernant le recrutement des praticiens hospitaliers et la gouvernance des hôpitaux. Comme les dispositifs de coopération renforcée, ils étaient pourtant au coeur du décloisonnement censé être porté par la loi de juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation de notre système de santé. Comment les professionnels peuvent-ils s'emparer des modalités d'exercice coordonné et de coopération locale, alors que celles-ci sont constamment remaniées ? Il en va de même pour les instances de gouvernance de l'hôpital : faute de vision globale, le Gouvernement s'enlise au milieu du gué. Aujourd'hui, alors même que la plupart des ordonnances concernées n'ont pas encore vu le jour, le Gouvernement sa majorité parlementaire accroît le flou en revenant sur des dispositifs non encore appliqués.

Le manque de sérieux dans la démarche est encore confirmé par le temps imparti pour l'examen de ce texte. À l'origine, cette proposition de loi, qui se veut pourtant ambitieuse et compte plus d'une trentaine d'articles, et dont certaines dispositions sont susceptibles de changer la gouvernance des hôpitaux, ne devait être discutée qu'en une demi-journée. Comprenant son erreur, le Gouvernement a demandé une modification de l'ordre du jour en dernière minute afin de permettre une demi-journée supplémentaire de débat. Ce changement contraint n'a cependant rien de satisfaisant. On nous demande de travailler dans la précipitation, sans pouvoir nous appuyer sur une enquête publique, pourtant nécessaire, pas plus que sur un avis du Conseil d'État, tout aussi nécessaire. Cette absence d'éléments justifierait à elle seule de siéger pendant plusieurs jours pour pallier les incohérences du texte et pour éviter l'adoption de mesures qui risquent de déstabiliser notre système de santé au plus mauvais moment. De fait, de l'Assemblée nationale au Sénat, cette proposition de loi, très succincte lorsqu'elle a été déposée par ses auteurs sur le bureau de la chambre basse, a d'ores et déjà fait l'objet d'un travail de réécriture extrêmement important, témoignant du grand manque de rigueur rédactionnelle et juridique de certains articles. Ce travail de réécriture a été aussi bien l'oeuvre du Gouvernement que des rapporteurs ; c'est dire l'impréparation de ce texte. Procéder ainsi est irresponsable et irrespectueux à l'égard du travail parlementaire, mais vis-à-vis des soignants. L'examen de cette proposition de loi aurait pu être l'occasion d'un débat et d'une réforme de la gouvernance hospitalière que la pandémie de la covid-19 a rendue plus que jamais nécessaire. Mais le choix du véhicule législatif, le temps très restreint imparti aux débats et l'engagement de la procédure accélérée nous empêchent de les mener sereinement. Il est ainsi flagrant que cette proposition de loi dépourvue de fil conducteur n'est qu'une tentative incomplète d'assemblage de mesures mal articulées entre elles. Il n'y a pas de vision globale de ce que devrait être notre système de santé rénové, pas de projet pour lui. Nous ne pouvons pourtant pas nous payer le luxe de voter des dispositions redondantes, insatisfaisantes, créant de nouvelles contraintes dont les conséquences n'ont pas été préalablement évaluées. Sur les trente-trois mesures que comporte le Ségur de la santé, seulement cinq sont reprises dans la proposition de loi. Elles ne font l'objet que de six des quarante-deux articles que comporte le texte après son passage à l'Assemblée nationale. C'est bien mince pour un texte censé traduire le volet non financier des conclusions du Ségur de la santé. L'article 10 de la proposition de loi correspond à la mesure 3 de ce Ségur, qui vise à mettre fin aux abus de l'intérim médical. La mesure 7 du Ségur, relative au renforcement du déploiement de la pratique avancée, permet à des infirmiers de réaliser des missions élargies par rapport à leur champ de compétences initial afin de répondre aux évolutions de l'organisation des soins. Cette mesure, qui était prévue à l'article 1, a été

vise à donner plus d'autonomie aux services des hôpitaux en matière de gestion et d'adaptation de leur organisation. Il s'agit de revenir à des unités plus concrètes, par exemple les services d'oncologie ou de cardiologie, plutôt que de renvoyer aux superstructures.

et les CSIRMT. La mesure 27 du Ségur visant à lutter contre les inégalités en santé, ou encore la mesure 31 visant à renforcer l'offre de soutien psychiatrique et psychologique, entre autres, sont absentes de la présente proposition de loi.

des mesures nécessaires dans une période où la santé mentale des Français est mise à mal par la pandémie de covid-19 et ses conséquences. Enfin, si les dispositions concernant les sages-femmes vont dans le bon sens, elles auraient pu faire l'objet d'un texte à part. Je conclurai mon intervention en soulignant que ce texte manque cruellement d'une vision globale. Nous n'avons pas suffisamment de recul pour nous prononcer sur des mesures dont les effets n'ont pour l'instant pas pu faire l'objet d'une quelconque évaluation. Nous ne pouvons pas légiférer sans visibilité. Par conséquent, nous demandons un renvoi du présent texte en commission afin de nous donner les moyens de l'examiner dans des délais plus appropriés et de disposer de davantage de visibilité quant aux ordonnances.

de légiférer en disposant d'une plus grande visibilité, notamment sur les ordonnances en cours. Cela reviendrait de plus à nier le travail important que nous sommes

même si nous connaissions le contenu des ordonnances en cours de publication, nous ne pourrions empiéter, par nos amendements, sur le champ de ces habilitations, en application de l'article 38 de la Constitution. Enfin, je doute qu'un délai supplémentaire nous permette de lever toutes les limites que nous reconnaissons à ce texte. En particulier, l'appréciation de son périmètre resterait

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons revêt par son titre de nombreux espoirs améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ». La crise sanitaire qui a frappé notre pays de plein fouet a mis en lumière les forces de notre système de soins, mais elle en a également relevé les faiblesses. Pendant la lente décrue de la première vague de contaminations, le Gouvernement a annoncé l'initiative intéressante d'un Ségur de la santé qui doit permettre une évolution tant attendue de l'organisation de notre La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui a pour objectif de traduire le versant non financier des conclusions du Ségur, enrichi des propositions du rapport Claris sur la gouvernance de l'hôpital. Toutefois, le véhicule législatif utilisé et la préparation concomitante d'ordonnances par le ministère de la santé compliquent l'exercice et nous privent d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État. Pour autant, la majorité du groupe RDSE, tout

travaillant de manière coordonnée et hors établissement. Cette disposition répond aux besoins d'une médecine plus coordonnée au bénéfice du patient, en ville comme à l'hôpital. La faible démographie médicale, mais aussi l'explosion des maladies chroniques, l'aspiration des jeunes à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que l'appétence pour l'exercice en équipe pluridisciplinaire, impliquent impliquent absolument et nécessairement l'évolution du champ des compétences des professionnels de santé. Nous aurons à examiner de nombreux amendements relatifs aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux. Certaines propositions vont seule philosophie doit nous guider : il faut améliorer et fluidifier le parcours du patient sans le détricoter. Le médecin généraliste est et doit en rester le pivot. Le Ségur a également mis en évidence l'existence, bien antérieure à la crise du covid, d'une perte d'attractivité des métiers de la santé. Les hôpitaux et les structures médico-sociales peinent d'ailleurs à recruter. La revalorisation légitime des salaires ne permettra pas, seule, d'y remédier. De bonnes conditions de travail, davantage d'effectifs dans les services, une gouvernance moins technocratique et plus médicalisée,

médicales publiques, privées ou associatives, et des freins à l'exercice d'un médecin sous différents statuts. Aussi, je proposerai d'y remédier en partie par la réintroduction de deux articles, dont l'article 14 , lequel, au-delà de la remise d'un rapport, permettra de ne pas enterrer trop précocement cette problématique. S'il est un sujet dont la crise a relevé les limites, c'est bien celui de la gouvernance des établissements. L'article 5 consacré à l'organisation interne restaure la fonction de chef de service non pas en opposition, mais en complémentarité de celle de chef de pôle. L'organisation des pôles doit absolument rester une possibilité pour chaque établissement. La création de chefs de service et de chefs de pôle adjoints améliorerait encore le fonctionnement de l'hôpital. Le groupe RDSE a déposé des amendements en ce sens. Comment parler d'organisation sans évoquer les GHT ? Installés à marche forcée, leur fonctionnement est hétérogène. S'il n'est pas souhaitable méritent d'être encouragés, sur la base du volontariat. L'article 9 de la proposition de loi ouvre le directoire de l'hôpital en prévoyant la possibilité pour le directeur de désigner des personnalités qualifiées. C'est à notre sens une bonne chose. Je regrette cependant l'exclusion des étudiants au sein de ce directoire. Je terminerai en évoquant les abus de l'intérim médical qui pénalisent lourdement, à la fois, les finances et le fonctionnement de l'hôpital. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Malgré la volonté exprimée en 2017 par le Gouvernement d'y mettre un terme, force est de constater que le problème Il est devenu urgent de mettre fin à ces pratiques que je qualifierais de scandaleuses, et de permettre enfin l'application du plafond des rémunérations. L'hôpital ne peut pas et ne doit pas être une zone de non-droit dans laquelle certains professionnels imposeraient des exigences financières déraisonnables. déraisonnables. Cette proposition de loi se présente comme un patchwork de mesures qui s'expliquent par le destin singulier de ce texte, pensé avant la crise sanitaire, puis saisi opportunément comme le moyen d'y intégrer quelques mesures du Ségur et tout ce qui n'entre pas dans le champ des ordonnances. Suffira-t-elle à satisfaire les attentes ? En tout état de cause, le groupe RDSE réservera son vote en fonction de l'évolution des discussions et il émet le voeu que les mesures consensuelles issues du Ségur et du rapport Claris puissent trouver une traduction législative.

Derrière les mots « simplification » et « confiance », il faut lire : « management public des hôpitaux et autonomie renforcée pour gérer l'austérité ». La proposition de loi de la députée Rist, qui est en réalité celle du Gouvernement, est pour le moins hétéroclite mais non dépourvue de cohérence puisqu'elle tend à l'affaiblissement du service public. Plutôt que d'investir massivement et durablement dans notre système de santé, ce texte propose de ronger les murs porteurs de l'hôpital. Après un Ségur raté, vous nous proposez une loi fourre-tout qui ne répond en rien aux attentes des soignants, ni même des usagers. Depuis trente ans, les politiques d'austérité ont entraîné la fermeture d'hôpitaux, de maternités, de centres de santé publique, de caisses d'assurance maladie. L'éloignement des services publics a créé une véritable rupture d'égalité, notamment pour les plus fragiles. À l'heure des débats sur le séparatisme, votre politique d'affaiblissement des services publics renforce le séparatisme financier qui met son argent au Luxembourg. Vous renforcez aussi le séparatisme économique qui licencie après avoir bénéficié de milliards d'aides publiques. Enfin, vous renforcez le séparatisme social de celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder aux soins. Cette proposition de loi donne l'illusion aux personnels hospitaliers qu'en contrepartie du renforcement de l'autonomie des hôpitaux, ils pourront dégager des économies suffisantes pour sortir des baisses des dotations. Quelle déception ! Quels mensonges ! Alors que certains services n'ont même plus les moyens d'acheter des couvertures pour les malades ni de renouveler le matériel vétuste, ce texte va aggraver la situation. En renforçant l'autonomie des hôpitaux, vous accélérez la mise en concurrence des établissements publics de santé entre eux, comme si celle avec les établissements privés lucratifs et non lucratifs ne suffisait pas. Vous créez une profession d'auxiliaire médical en pratique avancée. Vous avez certainement oublié l'activité professionnelle des infirmiers anesthésistes diplômés d'État, qui se livrent depuis de nombreuses années à un exercice de pratique avancée ! Je suis certaine que vous allez revoir votre copie et que vous allez les écouter ... Ne pensez-vous pas qu'il est temps, monsieur le ministre, de satisfaire les véritables besoins des personnels médicaux et paramédicaux ? C'est urgent et nécessaire. Arrêtez donc de présenter des lois qui ne sont que du bricolage à cinq sous ! Les personnels ont besoin de considération, de recrutements, de revalorisation salariale et d'amélioration de leurs conditions de travail. Telles sont les solutions pour Plutôt que de renforcer le pouvoir des chefs de service, il faut renforcer la démocratie sanitaire et garantir une meilleure représentation de l'ensemble des usagers, des personnels et étudiants en santé,

Votre dispositif anti-intérim se retourne contre les directeurs d'établissement, qui devront fermer des services plutôt que recourir à l'intérim s'ils veulent éviter les sanctions financières. financières. Il conviendrait au contraire de sanctionner les entreprises de travail temporaire qui ne respectent pas le plafond de rémunération. Nous proposons de rétablir les gardes de nuit, du week-end et des jours fériés, en indemnisant correctement les médecins qui effectuent ces astreintes.

la crise sanitaire a révélé les limites de notre système de santé. Elle nous a aussi permis de « reprendre » conscience du travail remarquable réalisé au quotidien par tous les professionnels qui participent à notre parcours de santé. Sommes-nous à la hauteur de leur investissement ? Répondons-nous clairement à leurs attentes légitimes ? Lancé en mai 2020, à l'issue du premier confinement, le Ségur de la santé a suscité beaucoup d'espoirs. Cet effort inédit est incontestablement une belle avancée. nombreux sont ceux qui nous disent avec amertume qu'il ne s'agissait pas du Ségur de la santé mais plutôt du Ségur de l'hôpital public Jour après jour, les parlementaires ont été et sont encore interpellés par des professionnels qui se retrouvent exclus des revalorisations sans en comprendre les raisons.

Aujourd'hui, nous examinons la proposition de loi de notre collègue députée, Mme Stéphanie Rist, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. objet de concrétiser les mesures non budgétaires du Ségur de la santé signé par les partenaires sociaux. Avant d'entrer dans le détail de l'examen du texte, je souhaite vous faire part de quelques remarques générales.

Cela promettait un examen au pas de course ! Je salue donc l'ouverture de la journée de jeudi pour examiner ce texte dans de bonnes conditions. Une proposition de loi ne permet ni étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Je le regrette, car ce texte porte

Les demandes d'entretiens et le nombre d'amendements proposés corroborent ce sentiment d'un manque total d'adhésion à cette proposition de loi. Je ne peux que regretter que les uns se sentent injustement écartés, quand les autres sont pour le moins déconcertés. garde, car nous ne sommes pas loin d'observer une réelle démotivation des professionnels. Je salue notre rapporteur, Alain Milon,

Enfin, cette proposition de loi se veut la traduction de la partie non budgétaire des conclusions du Ségur de la santé. Force est de constater qu'elle n'atteint pas cet objectif, puisque seulement cinq des trente-trois mesures du Ségur se retrouvaient dans le texte de commission de l'Assemblée nationale. J'entends les arguments de son auteure : « Nombre de mesures attendues par les professionnels de la santé relèvent du niveau réglementaire et des ordonnances prévues dans le cadre de la loi Ma santé 2022, et ne figurent donc pas dans ce texte. nous sommes en droit de nous interroger sur l'intitulé de cette proposition de loi. Vise-t-elle réellement à améliorer notre système de santé par la confiance et la simplification ? J'en doute. S'il y a urgence à redonner de l'attractivité aux carrières au sein des hôpitaux publics, les sentiments d'injustice et de frustration ne cessent de monter sur le terrain. Il faudra un jour y répondre Je m'arrête là pour les considérations générales, et j'en viens aux articles de la proposition de loi. Je commencerai par ce que je considère comme des avancées bienvenues. Il s'agit du chapitre II relatif à l'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux. Si les articles 2 et suivants n'engagent pas de révolution, ils sont autant de bouffées d'oxygène pour les professions concernées et surtout pour les patients. Il conviendrait d'amplifier ce mouvement. Aussi, une fois n'est pas coutume, je ne partage pas la position de notre rapporteur- qu'il me pardonne ! -sur l'article 2 B qui permettait aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un médecin spécialiste, sans pénaliser celles-ci en termes de remboursement des frais de soins Je ne crois pas que cette disposition induise une confusion dans la logique du parcours de soins coordonné, articulé autour du médecin traitant. C'est au contraire une mesure de simplification du parcours des patientes qui serait bienvenue, d'autant qu'elle est conforme à l'objet de la proposition Nous le savons, le temps de la grossesse est un temps à part dans la vie d'une femme. Les sages-femmes n'ont donc pas vocation à se substituer aux médecins. Aussi, dans un objectif de simplification du parcours de santé et d'un meilleur accès aux soins, j'ai déposé plusieurs amendements pour amplifier ce qui restait à l'état d'esquisse dans ce chapitre II. J'appelle cependant le ministre nous ne pouvons pas étendre indéfiniment le champ d'intervention de ces professionnels sans améliorer leur statut. Concernant la mesure phare portée initialement par l'article 1, je partage en tout point l'analyse de notre rapporteur. Introduire une nouvelle strate de professionnels de santé ne peut se faire sans l'assentiment des principaux concernés. Cela n'a pas été le cas. Dont acte. Le chapitre IV relatif à la gouvernance des établissements publics de santé suscite de vives réactions.

Dans la même dynamique, l'article 5 modifié par la commission est bienvenu tant la notion de « service » fait consensus chez les professionnels. Enfin, nous ne pouvons que souscrire à l'objectif d'associer davantage le personnel soignant à la gestion de l'hôpital, notamment par le biais de l'élaboration du projet médical, dont la finalité est de répondre aux besoins de santé de la population. Pour conclure, cette proposition de loi a fait naître des sentiments très ambivalents, oscillant entre l'espoir et la déception. Les mesures contenues dans le texte ne parviennent pas à se hisser à la hauteur des ambitions et des attentes bien légitimes de celles et ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en cette période particulièrement éprouvante. Le Sénat apporte un certain nombre d'améliorations salutaires. Aussi, le groupe Union Centriste votera favorablement le texte ainsi modifié.

À l'issue de son passage en commission au Sénat, neuf articles ont été supprimés. Le texte a un peu dégonflé, sans atteindre toutefois la taille usuelle d'une proposition de loi. Le rapporteur a procédé à un important travail de réécriture sur de nombreux sujets complexes et pourtant absolument essentiels pour notre système de santé. santé. Nous ne pouvons que déplorer le rejet de la motion de renvoi à la commission, qui aurait pu nous octroyer le temps nécessaire pour effectuer un travail à la hauteur des enjeux, en pleine conscience notamment des ordonnances en préparation. le choix d'un examen du texte bâclé. Or nous considérons que les soignants mobilisés depuis un an pour faire face aux différentes vagues de l'épidémie méritent mieux. Je m'attarderai brièvement sur quelques articles qui ont particulièrement retenu notre attention. L'article 1, supprimé par le rapporteur, visait à créer une profession médicale intermédiaire entre infirmiers et médecins sans en détailler les modalités techniques et juridiques. Face au mécontentement général, il est devenu une simple demande de rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération.

d'étendre les protocoles de coopération à tout le champ de l'exercice coordonné, alors même que les dispositions votées dans la loi Santé de 2019 sont encore à peine appliquées. Le chapitre II introduit quelques dispositions attendues et réclamées par les sages-femmes depuis longtemps. Même si

une unité pertinente dans la prise de décision, d'organisation et de mise en oeuvre de l'offre de soins, et que les réformes successives de l'hôpital les ont trop éloignés des instances décisionnelles. Pour autant, l'article 5 procède-t-il réellement à ce changement de cap ? ne le crois pas, et je doute que nous puissions promettre aux personnels hospitaliers le changement qu'ils attendent, si nous ne posons pas clairement la question de la répartition des compétences entre les pôles d'activités et les services. Dans la même logique, nous défendons une place plus importante donnée à la parole des personnels paramédicaux représentés au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. La gestion de la crise de la covid à l'hôpital a souvent permis de « mettre autour de la table » la direction, les médecins et les soignants, dans le cadre d'un travail collectif pour organiser la prise en charge. Les verrous financiers ne sont pas les seuls à être passés au second plan pendant cette crise : celui de la verticalité, souvent bureaucratique,

Pour cette raison, nous nous opposerons aux dispositions de l'article 6 qui prévoient la fusion de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT). Nous sommes convaincus qu'il faut au contraire conforter une plus grande autonomie de la CSIRMT, et par conséquent ne pas permettre une telle fusion.

Enfin, la proposition de loi s'achève sur un énième article décevant sur le handicap. Le Ségur de la santé n'a-t-il pas d'autres ambitions pour le secteur médico-social que la commande d'un rapport et l'instauration d'une plateforme en ligne venant s'ajouter à un numéro vert déjà en place et dont tout le monde s'accorde à dire qu'il ne remplit pas son rôle ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise du coronavirus aura eu un mérite celui d'avoir mis en lumière l'état d'extrême fragilité, pour ne pas dire de délabrement, dans lequel se trouvaient nos hôpitaux, conséquence d'un abandon délibéré des pouvoirs publics, qui ont considéré la santé des Français comme un luxe qu'il convenait de réduire au nom d'une gestion financière saine. Le résultat de l'approche prioritairement financière de la santé, nous le connaissons : le deuil des familles, la fatigue et la colère d'un personnel médical dont le courage ne suffit plus à encaisser la mutation du serment d'Hippocrate en discours d'hypocrite de la part de leurs ministres de tutelle successifs. Le mal ne se résume pas à l'état catastrophique dans lequel se débat l'hôpital public. Il frappe tous les domaines liés à la santé. Au manque de places, d'équipements et de personnels dans nos hôpitaux s'ajoutent la pénurie de médecins en ruralité, la suradministration, les étriqués et dépassés, la disparition de notre production nationale de produits pharmaceutiques- qu'il s'agisse des masques chirurgicaux, mais aussi des vaccins et des médicaments l'abandon par l'État des chercheurs et des entreprises innovantes, les restrictions budgétaires sans vision de long terme imposées par Bruxelles. Or, dans un pays qui se veut l'un des plus riches, des plus accueillants, des plus protecteurs, la santé des citoyens ne devrait pas être considérée d'abord comme un coût, mais comme un investissement. Ce texte est encore bien éloigné d'une telle perspective. Les leçons de la crise sanitaire, qui est loin d'être terminée, ne sont manifestement pas tirées. Se préparer au pire, pour éviter de le vivre ou de le revivre, n'est toujours pas à l'ordre du jour. Continuer de refuser le principe de précaution est une erreur, et refuser la souveraineté et donc l'indépendance sanitaire est une faute. Dans cette proposition de loi je retiendrai et soutiendrai néanmoins la revalorisation de la profession de sage-femme. En effet, les sages-femmes sont les garantes d'un accompagnement personnalisé optimal pour les femmes et les nouveau-nés. Elles mettent en place les meilleures conditions pour que se développe la natalité française, dans un contexte où l'on craint pour l'avenir. Elles suivent et rassurent les femmes pendant la grossesse, assurent l'accouchement et accompagnent la mère et l'enfant pour les soins de post-natalité. Je soutiendrai dans ce texte l'élargissement du périmètre de leur activité. Trop souvent considérées comme exerçant une profession paramédicale, les sages-femmes doivent pouvoir varier leurs prérogatives médicales et obtenir une rémunération à la hauteur de leur diplôme, de leur statut et surtout de leurs responsabilités. Cependant, le salaire ne fait pas tout, et il n'efface pas l'épuisement. Tout cela ne servira à rien si l'on n'augmente pas le nombre de sages-femmes. Le mouvement populaire « Une femme = une sage-femme » pointe l'insuffisance des effectifs qui conduit à une prise en charge des patientes insatisfaisante,

Dans l'ensemble, alors que tout devrait être revu de fond en comble, ce texte présenté dans la précipitation manque cruellement d'ambition. Pourtant, nous le savons, les économies d'hier nous coûtent très cher aujourd'hui, et pas seulement financièrement. Malgré ces insuffisances et devant l'urgence de la situation, je voterai ce texte.

et je voudrais saluer le rapporteur qui a oeuvré en ce sens. La création de l'exercice d'infirmier en pratique avancée, accessible après trois ans, est une bonne initiative.

privilégier le dispositif de pratique avancée, en incluant les infirmiers anesthésistes, comme le propose mon collègue Alain Marc. En revanche, nous devons mieux travailler avec les pharmaciens, qui contrôlent les ordonnances et conseillent les patients, qui sont des acteurs de premier plan en qui participent aux vaccinations et font des substitutions de médicaments, mais qui ne sont pas autorisés, pour l'instant, à prescrire un médicament pour les cystites, pas même un examen d'urine. Commençons par améliorer l'existant plutôt que de créer une nouvelle profession

des praticiens hospitaliers. En effet, il faut donner aux établissements la possibilité d'être plus réactifs en simplifiant les procédures trop lourdes. Il faut aussi revaloriser les salaires. L'article 5

associer le personnel, les internes et les paramédicaux au projet de l'hôpital. L'article 7 avait pour objet de renforcer l'intégration des GHT par le prisme des directions communes. Cela permettait, avec l'accord des élus locaux et des CME, de développer une vision cohérente du territoire. Cette direction commune entre établissements d'un même GHT me semble être la solution la plus efficace et la plus adaptée pour mettre en oeuvre un projet médical partagé avec l'établissement support, en veillant dans la mesure du possible à faire du département l'échelon préférentiel d'organisation du GHT. Je soutiendrai l'amendement de mon collègue Franck Menonville visant à renforcer le rôle des élus locaux au sein des conseils de surveillance. L'article 7 a pour objet la création d'un service d'accès aux soins non programmés qui aura pour tâche d'améliorer la demande de soins en amont des urgences, et de diriger les patients vers un professionnel de santé pour une consultation sans rendez-vous. Nous devons mettre en place ce dispositif sur l'ensemble du territoire.

vise à lutter contre les abus de l'intérim médical. Il faut savoir que les établissements sont dépendants de ce recours pour assurer la continuité des soins, notamment dans certaines spécialités.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout a été dit sur l'immense déception de la quasi-totalité des acteurs de santé quant à cette proposition de loi- après le Ségur, le rapport Claris, le mouvement social et surtout la crise sanitaire -, tant sur le fond que sur la méthode. Si nous saluons l'abandon de la création d'une profession médicale intermédiaire, il convient de rappeler que la reconnaissance et l'évolution attendues des compétences, en vue d'un décloisonnement des professions de santé,

Cette offre doit s'articuler et non se confondre ou entrer en concurrence avec les spécialisations infirmières en bloc opératoire, puériculture ou anesthésie, dont le champ de compétences et d'exercice comprend, de fait, celles requises pour la pratique avancée paramédicale. Dès lors, avec des moyens humains à la hauteur des besoins, l'effet sur l'efficience du temps médical aura un impact positif. La proposition de loi poursuit la lente mais nécessaire reconnaissance du métier de sage-femme, profession médicale à part entière, à compétences définies mais sous-déployées. II est temps de poursuivre l'élargissement du champ de compétences des sages-femmes à partir de leur coeur de métier, et de reconnaître leur place dans le parcours de soins, et le décloisonnement entre

C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires soutient les articles en ce sens et les enrichira. Rappelons que pour cette profession comme pour d'autres, le compte des accords du Ségur n'y est pas, ce qui justifie le mouvement social actuel.

il faut aussi améliorer rapidement les conditions d'exercice à l'hôpital, en recrutant massivement pour renouer avec le sens du travail bien fait, et permettre la réduction du temps de travail et du recours obligé aux heures supplémentaires. L'intérim reste parfois le seul moyen de maîtriser son temps. En attendant, l'injonction paradoxale entre continuité du service et soumission au chantage des sociétés intérimaires ne peut peser sur le seul directeur d'établissement. Autre axe de cette proposition de loi, la gouvernance acte le retour du service ou, du moins, sa réaffirmation après la contestation majoritaire de l'organisation par pôles.

l'hôpital reste largement médico-centré, vertical et descendant, loin des aspirations des jeunes générations de salariés qui, au-delà de salaires décents, aspirent à davantage de participation aux décisions. La gouvernance, élément essentiel de l'attractivité, attend toujours sa réforme en profondeur. La parole

la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification se veut la traduction législative des conclusions du Ségur de la santé, celles du moins qui ne relèvent pas du domaine budgétaire. À l'Assemblée nationale, ce texte a été profondément modifié, complété, amélioré pour que les attentes et les besoins du personnel médical et des patients soient mieux pris en compte. Ce texte, mes chers collègues, n'a pas pour objet de révolutionner l'organisation de notre système de santé. Il n'a pas non plus vocation à répondre à l'ensemble des difficultés que la crise sanitaire a mis en exergue. Il s'agit d'une pierre supplémentaire qui s'ajoute aux réformes déjà menées par le Gouvernement, et qui en appelle évidemment d'autres. En septembre 2018, le plan Ma santé 2022 prévoyait ainsi de transformer en profondeur notre système de santé. Cinq actions prioritaires étaient définies, parmi lesquelles l'accélération de la mise en place des communautés de médecins généralistes dans les territoires prioritaires et la création de postes d'assistants médicaux. Dans la foulée, et pour répondre à la mobilisation du personnel urgentiste, le pacte de refondation des urgences a permis d'affirmer la nécessité des services d'accès aux soins, de renforcer l'offre de consultations médicales sans rendez-vous, et de généraliser les parcours dédiés aux personnes âgées. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a assuré la mise en oeuvre des engagements budgétaires du Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, rappelons-le, ce sont des engagements sans précédent en faveur du monde médical et paramédical. C'est aussi la revalorisation des salaires du personnel des établissements de santé et des Ehpad. C'est un plan d'investissement de 19 milliards d'euros en faveur des établissements de santé. C'est enfin la poursuite des innovations organisationnelles et la promotion de la télémédecine. Mais la crise sanitaire a également révélé l'urgence de simplifier l'organisation de notre système de santé et le besoin de reconnaissance de tous les professionnels.

remodelé en commission des affaires sociales. Force est de constater qu'il reste bien peu de choses du texte initial. Certaines de ses dispositions ont toutefois fait l'unanimité, et nous saluons la volonté du rapporteur de les conserver. Le chapitre II prévoit ainsi d'élargir les compétences des sages-femmes en matière de prescription des arrêts de travail, ou de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles. Il en va de même pour les masseurs-kinésithérapeutes, qui verront leur faculté de prescription clarifiée. Nous nous réjouissons que ces revendications anciennes trouvent enfin leur place dans un texte de loi. Le chapitre IV, consacré à la gouvernance des établissements publics de santé, conserve également certaines dispositions importantes. L'article 5 réhabilite ainsi le rôle et la place du service au sein de l'hôpital. L'article 10 prévoit en outre de lutter contre les abus liés à l'intérim médical, qui grèvent les finances des établissements publics. L'article 14, enfin, inscrit dans la loi la création d'une plateforme numérique d'information et de services à destination des personnes handicapées, plateforme qui a été déployée en mai dernier et qui poursuivra sa montée en puissance. À l'inverse, certaines dispositions que nous pensions nécessaires ont été supprimées. Nous le regrettons et proposerons d'en rétablir quelques-unes. C'est le cas notamment de l'article 1 qui visait la remise d'un rapport consacré à la pratique avancée et aux protocoles de coopération. Cet article étant le fruit d'un compromis, nous proposerons de revenir sur sa suppression, tant il nous paraît essentiel d'avancer sur le sujet. L'article 4 tendait, quant à lui, à instaurer un cadre légal pour l'intervention individuelle de praticiens bénévoles dans les établissements publics de santé. Nous proposerons de réintégrer cette disposition en apportant un certain nombre de garanties concernant leur formation et leur encadrement. Nous proposerons par ailleurs de revenir sur la suppression de l'article 11 consacré à la création d'un projet managérial participatif à l'hôpital, article auquel nous proposons d'ajouter un volet numérique. Cet outil nous semble en effet aller dans le sens d'une meilleure gestion des hôpitaux et, donc, de la simplification de notre système de santé. Pour finir, nous proposerons d'inscrire dans la loi l'importance de mettre en place, au sein des GHT, un système d'information convergent et interopérable,

d'émailler l'examen de cette proposition de loi, constatant enfin l'usage très généreux qui a été fait de l'article 45 de la Constitution, le groupe RDPI réservera son vote en l'absence d'avancées significatives. La parole

Monsieur le ministre, alors que vous nous aviez habitués à présenter des textes qui n'avaient pas toujours les moyens de leurs ambitions, nous avons découvert avec étonnement un texte qui n'avait pas les ambitions de son titre Le Ségur de la santé, qui a eu lieu entre mai et juillet derniers, s'annonçait pourtant prometteur. Or cette proposition de loi, présentée comme la traduction législative des mesures issues de cet accord qui ne relèvent pas du domaine budgétaire, est plus que décevante. Nous ne pouvons que que le regretter. La crise sanitaire a de nouveau illustré la lourde tâche qui incombe quotidiennement aux professionnels de santé. Il est devenu urgent de revaloriser ces professions à la hauteur de la responsabilité qui est la leur. Toutes les voies possibles ont été explorées, afin de recueillir le maximum de points de vue et de témoignages : concertations, groupes de travail, consultations en ligne. Plusieurs thématiques avaient été déterminées à l'avance, afin de déterminer les objectifs et les solutions proposées pour répondre aux malaises des personnels soignants. À l'image du grand débat national, la méthode utilisée lors de ce Ségur était annonciatrice des limites qui seraient atteintes lors de la traduction législative de ces enjeux primordiaux. En effet, monsieur le ministre, nous sommes plusieurs dans cet hémicycle à vous avoir alerté sur les conséquences prévisibles d'une limitation du Ségur de la santé à certaines professions de santé et, en particulier, sur le fait d'exclure les professions de santé libérales. À l'image de son cheminement, cette proposition de loi est hospitalo-centrée. Elle ne saisit pas l'essence même des difficultés rencontrées quotidiennement par nos concitoyens en matière d'accès aux soins. Notre système de santé est un tout. On ne peut pas prétendre le simplifier en se limitant à certaines professions. professions. Cela crée au minimum de l'incompréhension et provoque, dans le pire des cas, un profond sentiment d'iniquité et de colère. Je reviendrai également sur le vecteur législatif utilisé pour traduire les conclusions du Ségur. Est-ce de l'impréparation ? C'est peut-être un euphémisme quand on sait que ce texte a été déposé une première fois, puis retiré faute de cohérence et de solutions, avant d'être à nouveau redéposé, alors que les premières interrogations n'avaient toujours pas trouvé de réponses satisfaisantes. Je m'interroge également sur la pertinence d'aborder une thématique de cette ampleur par le prisme d'une proposition de loi. Un projet de loi semblait bien plus adapté et, surtout, davantage à la hauteur de l'enjeu que représentent les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et l'ensemble de nos concitoyens en matière d'accès aux soins. La simplification est une attente, c'est vrai. La confiance, elle, se mérite ! En fait, je doute profondément de la méthode choisie par le Gouvernement pour aborder ce dossier auquel nous sommes évidemment très attachés, et à propos duquel les attentes étaient fortes. Que dire d'un texte qui fait référence à des ordonnances qui, à ce jour, n'ont pas été publiées ? Que dire d'un texte sur lequel, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi, l'avis du Conseil d'État n'a pas été sollicité ? Vous avez déjà répondu à cette dernière question : le Gouvernement a souhaité mieux valoriser l'initiative parlementaire en privilégiant cette méthode de travail. Il est vrai qu'un des travers de ce quinquennat a souvent été de vouloir abaisser le rôle du Parlement. Et pourtant, j'ai du mal à me faire à l'idée que cette proposition de loi marquerait un regain d'intérêt de la part de l'exécutif vis-à-vis du pouvoir législatif. Monsieur le ministre, les avis exprimés par l'ensemble de mes collègues, sur de nombreuses travées de cette assemblée, sont révélateurs de la profonde déception qui est la nôtre concernant ce texte. Son champ d'action très limité nous a empêchés d'aborder de nombreuses thématiques qui semblaient pourtant prioritaires et urgentes. Bon nombre de catégories de professionnels de santé ne comprendront pas qu'après une loi Ma santé 2022 en demi-teinte, cette proposition de loi se concentre principalement sur la médecine hospitalière. Pour autant, le groupe Les Républicains a souhaité travailler sur ce texte et l'enrichir. de cette ambition d'améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, nous avions perçu une volonté forte de faire en sorte que le parcours des patients soit plus simple, et ce avec une qualité de soins identique sur l'ensemble du territoire, nous aurions pu nous y retrouver. Hélas, ce texte ne règle pas grand-chose. Les professionnels de santé sont désabusés. Plus qu'une faute politique, c'est une faute morale que commet l'exécutif en proposant un texte si peu ambitieux et si peu convaincant. Le temps long, si cher à notre Haute Assemblée, saura vous le rappeler : vous aviez vu, vous aviez su, mais en définitive, vous auriez dû Et puisque la confiance figure dans l'intitulé de ce texte, monsieur le ministre, je profite du temps de parole qui m'est donné pour vous demander si vous entendez publier rapidement le décret d'application de la mesure votée sur l'initiative du Sénat dans la loi Santé de 2019, qui impose aux internes en médecine de troisième année une période de professionnalisation d'au moins six mois en zone sous-dotée.

depuis de très nombreuses années, l'hôpital public est en souffrance : le manque de moyens et son corollaire, la fermeture de postes et de lits, la reconnaissance salariale insuffisante complexité de son organisation entraînent une carence d'attractivité chronique de nos hôpitaux. Et pourtant, la réponse des personnels à la pandémie a été, et est encore, remarquable et admirable. Dans ce contexte particulier, alors que le Ségur de la santé et le rapport extrêmement documenté et riche en préconisations du professeur Claris ont fait naître un certain espoir, nous examinons une proposition de loi qui, malgré son titre attractif, ne suscite que déception et frustration. Comme l'ont déjà souligné mes collègues, la forme interroge. Cette proposition de loi, en ne reprenant que peu des dispositions du Ségur de la santé- cinq sur trente-trois -, ne répond en rien aux attentes du monde médical et hospitalier. Pire encore, elle crée une insécurité juridique et des incompréhensions.

dont beaucoup ont été supprimés ou entièrement réécrits dès son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, preuve de son impréparation ! Sur le fond, cette proposition de loi s'attaque-t-elle véritablement au problème de l'attractivité de nos hôpitaux publics ? Tient-elle compte des remontées de terrain et de la vraie vie des personnels et des usagers ? Absolument pas ! Ce texte balaie, au contraire, un nombre important de sujets sans apporter de réponse de fond ou de vision globale. Il ne fait qu'effleurer les principales préoccupations du monde hospitalier. Loin de renforcer l'attractivité des carrières hospitalières et de valoriser les personnels soignants, le texte comporte même, sous couvert de simplification, des mesures contreproductives, tels que le bénévolat individuel ou la possibilité pour un directeur de GHT de créer un poste de praticien hospitalier. La création d'un service d'accès au soin aurait également mérité un travail plus approfondi entre l'hôpital et la médecine de ville, en particulier avec les maisons pluridisciplinaires de santé ou les établissements de soins primaires.

Certes, il existe quelques propositions intéressantes. Je pense en particulier aux mesures concernant les sages-femmes ou les kinésithérapeutes, mais l'ensemble inspire un sentiment de déception et de frustration, qui risque de démobiliser l'ensemble du personnel hospitalier.

de cette proposition de loi était de poursuivre ce que le plan Ma santé 2022 a engagé à travers la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il paraissait en effet nécessaire de simplifier les protocoles permettant aux acteurs de santé de coopérer, en déléguant certaines tâches notamment, mais aussi de faciliter le recrutement de praticiens hospitaliers, en particulier dans les GHT, afin de mieux prendre en charge les patients et d'améliorer l'offre de soins. puis la crise sanitaire est intervenue. Elle a souligné le rôle essentiel de nos médecins et soignants. Dans ses conclusions présentées en juillet 2020, le Ségur de la santé a prévu les revalorisations salariales qu'attendaient ces personnels, de la sécurité sociale que nous avons voté en fin d'année. Si d'autres mesures, qui ne relèvent pas du domaine budgétaire, sont pour partie reprises dans le texte que nous examinons aujourd'hui,

bien que ces derniers soient par nature des établissements du service public hospitalier accomplissant les mêmes missions et ayant les mêmes devoirs vis-à-vis des usagers que l'hôpital public. Ainsi, les médecins du secteur privé non lucratif ont été exclus des dispositifs de revalorisation salariale. Le différentiel de rémunération est tel qu'il se traduit par une perte d'attractivité des postes de médecins dans les Espic. Cela va même plus loin puisque, aujourd'hui encore, alors que dans les établissements publics les praticiens peuvent exercer une activité libérale, avec dépassements d'honoraires et reste à charge pour les patients, les médecins exerçant dans les Espic n'en ont pas

Des mesures simples, telles que celles que nous proposons, peuvent renforcer l'attractivité de l'ensemble de nos hôpitaux, quel que soit leur statut juridique, d'autant que les uns et les autres permettent d'amplifier l'offre de soins sur nos territoires. Nos hôpitaux fonctionnent bien souvent de façon parfaitement complémentaire, les usagers ne faisant aucune différence entre les diverses structures. Si l'on veut favoriser l'attractivité des hôpitaux publics et des Espic, commençons par harmoniser les conditions de travail. Alors que nous évoquons la nécessité de mettre en place un exercice coordonné des pratiques et la complémentarité des acteurs du soin, une telle harmonisation de l'exercice mixte me paraît indispensable.

en cette fin d'après-midi, on nous demande d'examiner brièvement une proposition de loi qui se voudrait la traduction du Ségur de la santé. Les défis sont de taille et nous appellent à redoubler d'efforts. À l'issue du Ségur,

lutter avec une énergie nouvelle contre les inégalités de santé, de donner plus de voix aux soignants dans la gouvernance des établissements de santé, de mieux tenir compte des enjeux environnementaux, de mettre le numérique au service de la santé de tous, et tout cela dans l'intérêt supérieur des patients et de leur santé ». La proposition de loi que nous examinons en procédure accélérée répond-elle à cet objectif de traduire dans notre droit les objectifs du Ségur ? Malheureusement non. Ce texte ne répond pas à son ambition initiale, et les mesures proposées pour l'hôpital public restent largement insuffisantes. La pandémie a pourtant mis en exergue les dysfonctionnements de l'hôpital et l'exaspération des soignants, qui sont épuisés et se sentent insuffisamment pris en considération. Nos infrastructures sont souvent vétustes, et le nombre de lits reste insuffisant depuis le début de la pandémie. Les sujets essentiels, comme la formation ou l'organisation de la médecine de ville, sont complètement éludés. Concernant l'aspect financier, nous sommes tous conscients de la nécessité de revaloriser les salaires des personnels médicaux et paramédicaux. Il est impératif de fixer des salaires décents au regard des responsabilités et de l'engagement des soignants. outre, il est urgent de favoriser l'installation des médecins sur l'ensemble du territoire et de résorber les déserts médicaux. Mais cette traduction du Ségur de la santé ne propose aucune mesure forte. En ma qualité de médecin et de parlementaire, je regrette ce décalage entre les mesures annoncées lors du Ségur de la santé et cette proposition de loi aux mesurettes disparates. Monsieur le ministre, ce texte aurait pu être l'occasion d'une vraie réforme, mais son contenu et la procédure accélérée ont considérablement amoindri l'ambition de ses auteurs. De plus, le périmètre de la proposition de loi initiale et les règles en matière de recevabilité des amendements, qui découlent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n'ont pas permis au Sénat d'enrichir le texte, afin de répondre aux attentes des professionnels de santé et des patients. Malgré tout, le rapporteur et les commissaires des affaires sociales ont pu le remanier et l'améliorer. Dix articles sur trente-sept ont été supprimés, notamment l'article 1qui, dans sa version initiale, prévoyait la création d'une « profession médicale intermédiaire », en d'autres termes un médecin au rabais. Faisant l'unanimité contre elle, cette proposition a été abandonnée dès son examen par l'Assemblée nationale pour être remplacée par une disposition prévoyant la remise d'un rapport au Parlement dans un délai d'un an, qui a été supprimée à son tour. L'article prévoyant l'intervention de bénévoles à titre individuel dans les établissements publics et privés de santé en dehors du cadre associatif Les compétences des sages-femmes en matière de prescriptions d'arrêt de travail ou d'examens de dépistage et de traitement ont été élargies. Je me réjouis aussi que la lutte contre le recours abusif à l'intérim médical ait été améliorée. Les attentes des soignants et des Français sont importantes. Ce texte improvisé et insuffisant, dont nous ne saisissons pas les objectifs, risque de les décevoir une nouvelle fois. Néanmoins, nous allons tâcher d'améliorer cette proposition de loi dans un délai extrêmement court au regard des enjeux.

Madame la sénatrice Imbert, vous m'avez posé une question sur le renforcement de l'attractivité des zones sous-denses pour favoriser l'appropriation des futurs métiers. Vous avez notamment parlé de la maîtrise de stage ambulatoire. Nous visons deux objectifs, qui sont pour moi indissociables : l'augmentation du nombre de maîtres de stage

sur l'état d'esprit qui règne depuis plus de dix ans dans nos établissements de santé. Je ne dis pas pour autant que la réforme était mauvaise. Je dis simplement que les transformations sont nécessaires au bout d'un certain temps, au terme d'un certain cycle, quand on se rend compte que

binôme. Je crois profondément qu'en donnant la possibilité aux uns et aux autres de modifier leur gouvernance interne, on apporte une solution à beaucoup de problèmes. L'un des maux qui ronge l'hôpital- il n'en a pas été question lors de la discussion générale -, ce sont les conflits interpersonnels.

Théophile. Initialement, l'article 1 visait à établir un cadre législatif pour une nouvelle profession intermédiaire. Après avoir repris l'une des conclusions du Ségur de manière peut-être prématurée, nos collègues députés ont transformé cet article en une demande de rapport, contribuer au déploiement de l'exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération. Il est évident que la situation actuelle ne répond pas aux besoins d'évolution en compétences des professionnels de santé. C'est pourquoi ce rapport nous semble essentiel pour poursuivre la montée en puissance des leviers définis dans le plan Ma santé 2022. En effet, alors que l'accès aux soins sur le territoire est hétérogène, alors que les protocoles de coopération n'ont eu qu'un essor limité depuis 2009 et que la loi de juillet 2019 a récemment refondu leur cadre juridique, alors qu'un rapport de notre rapporteur soulignait en 2014 le besoin d'une montée en compétences et la nécessité de créer des professions intermédiaires, peu d'analyses existent sur la situation actuelle et sur ses limites On connaît le sort généralement réservé aux demandes de rapport dans cette assemblée, mais il me semblerait dommage de se priver d'éléments analytiques, alors même que c'est précisément, selon la commission, ce qui faisait défaut dans cette proposition de loi. En complément à l'occasion du Ségur, ce rapport permettra une analyse raisonnée et exhaustive de la situation actuelle, qui contribuera à répondre efficacement au besoin de simplification du système de santé. Pour toutes ces raisons, l'article 1 nous semble avoir toute sa place dans ce texte ; c'est pourquoi nous proposons

la portée de cet article est trop limitée au regard des enjeux réels de revalorisation des métiers de santé. Cette demande de rapport n'a pas sa place dans la loi, dans un article 1qui tend à en faire une disposition phare de ce texte.

de dispositifs n'ayant pas atteint leur pleine portée ou ayant fait l'objet de réformes récentes. Les premiers infirmiers en pratique avancée ont été diplômés en juillet 2019 et ils sont actuellement au nombre de 549.

J'entends et respecte, évidemment, les arguments du rapporteur et de la commission. Je ne vais pas revenir sur le fond de cette notion de profession médicale intermédiaire. Il ne s'agit certainement pas de médecins au rabais- l'enjeu n'est absolument pas là, et

vous », et non pas la députée qui a écrit cette proposition de loi. Au moins, c'est très clair ! Et vous avez missionné des représentants d'institutions de notre système de soins pour mener une réflexion à ce sujet. Très bien

de détermination dans notre système de santé, celle d'infirmier en pratique avancée et celle d'assistant médical ; dans les deux cas, c'est le cadre conventionnel qui est en train de travailler- vous suivez ces travaux de près -aux conditions d'émergence de ces professions, et c'est très bien comme ça. Je suivrai donc la position de la commission.

Cet amendement vise à permettre la constitution d'équipes coordonnées de soins autour du patient. L'idée est simplement d'accorder une reconnaissance à ces équipes de soins naturellement formées autour des patients et choisies par eux et de permettre aux professionnels de santé de se coordonner de manière souple et simple, sans avoir à créer de structure associative.

les conclusions de la mission pilotée par Nicole Notat sur le Ségur de la santé ont mis en exergue le besoin de développer des outils simples, notamment numériques, pour faciliter cette coopération. Il me semble toutefois que la définition de l'équipe de soins des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique est déjà relativement souple, puisqu'elle vise tout « ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte

ont en effet des compétences qui sont validées par des formations dont le cahier des charges- je le rappelle -est réglementé. Elles exercent déjà régulièrement ces compétences aux côtés des professionnels de santé. C'est d'ailleurs pour ces motifs que la Haute Autorité de santé a récemment recommandé

contre le VIH et sur le rapport dressé par la Cour des comptes, qui avait mené, à la demande du Sénat, une enquête sur les évolutions majeures de la politique de prévention et de prise en charge depuis 2010. La Cour recommandait une montée en charge, s'agissant notamment de mieux associer les associations agréées qui ont une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades. Quel est l'avis de la commission ? de la commission ? Cet amendement vise à étendre les protocoles de coopération entre professionnels de santé à des associations d'usagers du système de santé pour des activités de dépistage, de prévention et de diagnostic. L'idée est intéressante à l'heure du patient expert, ou pour reconnaître l'implication de ces associations. Toutefois, parce qu'il y a un « toutefois », il me semble que la mesure proposée conduit à assimiler ces acteurs à des professionnels de santé en en faisant des acteurs à part entière de protocoles de coopération.

en intégrant la profession réglementée des infirmiers anesthésistes dans le dispositif législatif existant. Cette profession ancienne, dont l'apport essentiel au système de santé est très largement démontré, durant la pandémie actuelle comme à chaque crise sanitaire ou événement exceptionnel d'ampleur,

Cet amendement vise à rattraper un oubli et à reconnaître ces professionnels de santé et leur pratique historique, essentiels en temps de crise comme au quotidien, tout en produisant un gain d'efficience pour notre système de santé.

sur l'engagement du Sénat pour que cet amendement soit voté et pour que soit réaffirmée la place effective qu'ils occupent au sein de notre système de santé. L'activité professionnelle des IADE constitue constitue depuis de nombreuses années un exercice paramédical avancé. Les infirmiers et infirmières anesthésistes bénéficient d'une formation et sont reconnus par leurs pairs, au niveau international, comme des professionnels en pratique avancée. La pandémie de covid-19 a démontré, s'il le fallait encore, l'utilité de leur polyvalence et la pertinence de leur modèle.

Cette qualification leur reconnaît une expertise technique dans un champ de compétences pluridisciplinaire qui regroupe l'anesthésie, la réanimation, les soins d'urgence et la prise en charge de la douleur aiguë et chronique. L'évolution défendue par les auteurs

liées à l'absence de valorisation de cette spécialisation ainsi qu'au projet de création d'un statut d'infirmier en pratique avancée dans le domaine des urgences, empiétant sur leur champ de compétences. Ces inquiétudes quant à une fragilisation de la profession d'IADE sont partagées par la société savante des anesthésistes réanimateurs, qui souligne le rôle essentiel des infirmiers anesthésistes et considère que, de fait, ils exercent déjà en pratique avancée, en autonomie déléguée aux côtés des médecins. Il serait intéressant,

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Les IPA ont vocation à se voir confier des missions vraiment transversales- consultations, interventions dans des structures très variées -, qui ne sont pas directement liées à une spécialité médicale, ce qui n'est pas le cas des IADE. Ceux-ci, je le répète, sont spécialisés dans le domaine des soins anesthésiques.

Une meilleure qualification des professionnels intervenant dans la prise en charge et le suivi des patients dans le cadre d'une prescription d'activité physique adaptée serait opportune, mais je doute que cela passe par la création d'une nouvelle profession de santé.

Le développement des protocoles de coopération est un levier majeur pour libérer du temps médical dans tous les territoires et, ainsi, adapter l'offre de soins à la demande. Il ne faudrait cependant pas perdre de vue la nécessité d'une réflexion globale sur les compétences des professionnels toujours dans la même perspective, de libérer du temps médical pour répondre à la demande de soins de nos concitoyens dans tous les territoires. C'est pourquoi je salue le travail sur cet article de la commission des affaires sociales, qui a rétabli les dispositions de la loi Santé de 2019 qui n'ont jamais été appliquées à ce jour. Il est important que cette possibilité soit offerte à tous les professionnels de santé travaillant en équipe, et non aux seules équipes hospitalières. Toutefois, je ne puis m'empêcher d'observer que, en dépit de notre activisme législatif collectif, les constats demeurent inchangés les inégalités territoriales dans l'accès aux soins s'accroissent et constituent une potentielle bombe à retardement. Il est donc dommage que cette proposition de loi ne permette pas de déployer des mesures plus ambitieuses. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, que j'ai l'honneur de présider, a formulé à plusieurs reprises des propositions afin de résorber les inégalités d'accès aux soins. Je souhaite que nous puissions collectivement avancer sur ce chemin et continuer à travailler sur d'autres dossiers essentiels, comme la régulation de l'offre de soins, la gouvernance des agences régionales de santé ou la télémédecine. décomplexification, permettrait de renforcer la dimension territoriale de la politique de santé. En attendant, nous devrons nous contenter de ce texte. La parole

dans nos réflexions le fait que le secteur privé participe, dans notre pays, au service public de l'hospitalisation et de la prise en charge médicale. Il est donc indispensable qu'un certain nombre d'améliorations soient aussi apportées dans le secteur privé.

Bernard Bonne. Le dispositif prévu à l'article 1 permet à des professionnels de santé exerçant au sein d'établissements médico-sociaux publics ou privés d'élaborer des protocoles locaux de coopération interprofessionnelle. Il autorise par conséquent des non-médecins à réaliser des actes médicaux qui relèveraient, hors de ce cadre, de l'exercice illégal de la médecine. Cet exercice dérogatoire, qui ne prévoit aucune relecture par une instance extérieure, pourrait remettre en cause la qualité des soins et la sécurité des patients et faire prendre aux professionnels de santé qui s'engageraient dans de tels protocoles une responsabilité considérable.

levait pas toutes les interrogations des professionnels de santé. Il serait toutefois dommage de priver totalement les équipes ambulatoires ou médico-sociales de la possibilité d'organiser des délégations d'actes, alors que la loi

Néanmoins, la dimension géographique et, au fond, la proximité de l'offre de soins sont déterminantes pour une prise en charge de qualité. Dans les départements ruraux, qui sont souvent des déserts médicaux, le temps de trajet entre le domicile et l'établissement de santé le plus proche influe directement sur le bien-être des citoyens et l'attractivité des territoires. Pour autant, l'offre de soins s'amenuise dans les territoires ruraux, plus particulièrement dans les territoires de montagne. À titre d'exemple, je citerai, dans les Hautes-Alpes, la fermeture du service des urgences de l'hôpital d'Embrun, le manque d'effectifs chronique dans les hôpitaux de Gap et de Briançon et la diminution importante de la population médicale. C'est pourquoi le maillage territorial de l'offre de soins doit être le dénominateur commun de tous les protocoles de coopération. Ces derniers doivent être le moyen non pas de mutualiser des services ou de fermer des unités, comme c'est le cas dans mon département, mais bien d'adapter l'offre de soins à un territoire donné.

Imbert, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié . Les protocoles de coopération permettent d'innover dans le parcours de soins et de répondre au mieux aux attentes des populations. De telles possibilités, élargies aux équipes de soins primaires, aux communautés professionnelles territoriales de santé, et aux établissements sociaux et médico-sociaux, les ESMS, par cette proposition de loi, doivent être ouvertes à d'autres structures accueillant des publics rencontrant des besoins spécifiques. Certains centres de santé, y compris ceux qui sont créés dans le cadre des expérimentations mentionnées à l'article L. 162-31-1 du code de la santé publique, font déjà le pari d'une approche adaptée aux populations qui les fréquentent. Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les Cegidd, qui concentrent des publics particulièrement exposés aux risques de contamination par les infections sexuellement transmissibles, doivent aussi pouvoir moduler leurs modalités d'accueil et d'accompagnement. Enfin, de nombreuses associations accueillent des professionnels de santé dans le cadre de leurs activités ; de fait, elles devraient être concernées par ces dispositifs et par les avantages qu'ils offrent. La parole

Quel est l'avis de la commission ?

mentionne explicitement les centres de santé, au titre de l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique relatif aux équipes de soins primaires. Par ailleurs, il existe également un protocole national de coopération qui est en cours d'instruction devant la Haute Autorité de santé. Il permettra par exemple aux Cegidd d'adapter leurs modalités d'accueil et d'accompagnement, comme vous le souhaitez. Enfin, il me paraît prématuré d'étendre cette possibilité aux associations agréées en dehors des cadres d'organisation susvisés par les textes de loi. C'est la raison

En effet, de plus en plus de protocoles nationaux sont communs aux professionnels de santé et aux professionnels du médico-social. Il est donc important le secrétariat d'État chargé du handicap soit intégré à la conception des protocoles. Le Comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de proposer la liste des protocoles nationaux de coopération à élaborer et à déployer sur l'ensemble du territoire et d'apporter un appui aux professionnels de santé dans l'élaboration de ces protocoles. Il est essentiel, puisqu'il contribue, entre autres, à élargir l'offre de soins dispensés et à améliorer les parcours de soins en déléguant à des personnels paramédicaux certaines activités jusqu'alors exercées uniquement par des médecins. Ce comité, rappelons-le, est composé de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels et les ordres des professions concernées sont associés aux travaux de ce comité. Le présent article prévoit d'intégrer à ce comité l'Union nationale des professions de santé, l'UNPS, qui regroupe vingt-deux organisations syndicales et professionnelles de santé en exercice libéral. L'UNPS n'est pas issue des élections professionnelles, comme le sont les unions régionales des professionnels de santé libéraux. Il s'agit d'une association suprasyndicale, dont les représentants sont désignés par les syndicats appartenant à l'UNPS. Il faut noter que plusieurs syndicats de professionnels de santé n'acceptent pas de confier à l'UNPS la mission de parler en leur nom. C'est pour cette raison que nous proposons un amendement de suppression de cet article. Quel

je ne vois pas d'obstacle à ce qu'une organisation comme l'UNPS, représentant, au niveau institutionnel, les acteurs libéraux, soit associée aux réflexions sur les protocoles de coopération.

afin de renforcer la lutte contre le tabagisme et d'améliorer les taux de morbidité et de mortalité des personnes accoutumées au tabac. La parole est

de la commission ? Ces nouvelles prérogatives me paraissent déjà incluses dans la mission générale de conseil des pharmaciens et dans les avancées actées par la loi Santé de juillet 2019 celle-ci a autorisé les pharmaciens, dans le cadre de protocoles inscrits dans un exercice coordonné, à délivrer pour certaines pathologies des médicaments dont la liste est fixée par arrêté,

du code de la santé publique prévoit déjà la possibilité pour les Ehpad de conventionner avec un pharmacien d'officine référent pour l'établissement qui concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. L'amendement étant satisfait, j'en demande le retrait. Quel est l'avis

nous proposons de reconnaître la place des sages-femmes dans les équipes de soins primaires. En effet, les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic des pathologies effectuées par les sages-femmes les positionnent comme praticienne de premier recours en soins primaires pour la santé des femmes. Ces professionnels sont donc au coeur du dispositif permettant à la patiente d'être au centre du parcours de santé. Cette place dans le système de santé français nécessite selon nous d'être clairement identifiée dans la loi. Un parcours de santé se définit comme la trajectoire globale des patients et usagers dans leur territoire, avec une attention particulière portée à la personne et à ses choix. Le parcours de santé des femmes est, quant à lui, l'organisation de la prise en charge globale et continue de celles-ci au plus proche de leur lieu de vie ou de travail. La lisibilité, l'accessibilité et la fluidité du parcours de santé s'appuient sur la qualité de l'information des conditions d'accueil et d'accompagnement de la femme tout au long de sa vie. Tous ces arguments plaident en faveur de la reconnaissance des sages-femmes dans les équipes de soins primaires. Cette mesure rejoint- une fois n'est pas coutume ! -la philosophie du plan Ma santé 2022, en élargissant les compétences des sages-femmes. Pour moi, comme pour l'ensemble des membres de mon groupe, cet amendement tend à s'inscrire dans la continuité des articles précédents visant à améliorer l'attractivité de cette profession, en travaillant sur la valorisation et la reconnaissance du métier. Mes chers collègues, cela fait plusieurs mois que les sages-femmes se mobilisent

: La parole est à M. Jean-François Longeot. Les soins dits « de premier recours », tels que les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic, de dispensation et d'administration des médicaments contribuent à pallier le manque de médecins et à assurer un meilleur accès aux soins des Français sur l'ensemble du territoire. Ces soins sont la plupart du temps administrés par les sages-femmes, praticiennes de premier recours pour la santé des femmes. Cependant, leurs compétences restent peu connues des patientes et d'autres professionnels de santé. Le présent amendement vise donc à reconnaître officiellement la contribution des sages-femmes à ces soins de premiers recours, contribution qui nécessite d'être clairement identifiée dans la loi. Quel est l'avis de la commission ? La rédaction de la commission ? La rédaction de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique sur les soins de premiers recours n'exclut pas les sages-femmes. soins découle par ailleurs de leurs missions, qui sont définies par les articles L. 4151-1 et suivants du code de la santé publique. Réaffirmer ce principe, comme le fait l'amendement n° 48 rectifié , aurait donc peu de portée.

définissent les compétences des sages-femmes et prévoient que ces dernières sont tenues d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique, ce qui est le cas en cas de suspicion d'infection par une Pour la sécurité des patientes, la prescription d'un traitement curatif doit relever du médecin, seul professionnel à disposer de la compétence pour prescrire un traitement curatif et à en assumer les conséquences. Quel est l'avis de la commission ? L'article

le champ au domaine de la prévention- les examens de dépistage des IST pour la femme et son partenaire -, en excluant le volet curatif, à savoir le traitement des IST chez les partenaires.

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise que les sages-femmes peuvent prescrire des dispositifs médicaux et des médicaments, selon une liste fixée par arrêté, ainsi que « les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession

encore, des sages-femmes. L'approche préventive des complications de la grossesse et des risques psychosociaux repose sur la création d'une relation de confiance entre futurs parents et professionnels de santé. Or ceux-ci sont souvent nombreux et ils sont surtout multiples, au cours du suivi, ce qui suscite parfois de la confusion et une perte de confiance. Il est donc nécessaire de coordonner les interventions sans les multiplier, afin d'assurer la cohérence et la gradation des propositions, adaptées aux besoins et à la temporalité des parents. Un référent de parcours doit être identifié dès le début de la grossesse, soit, lors de l'inscription, au sein de la maternité, soit, en ville, au moment de la découverte de la grossesse. Cette identification doit s'accompagner de la possibilité, pour les parents, de s'adresser à la sage-femme ou au maïeuticien qu'ils ont choisi comme référent, afin de poursuivre et de personnaliser l'accompagnement.

qui tiendra à jour le dossier médical. Il s'agit d'une évolution souhaitable du modèle périnatal français, visant à mieux répondre aux besoins et aux attentes des femmes et des professionnels. L'amendement n° 101,

Pour ce faire, il faut renforcer la coordination du parcours des femmes enceintes. En effet, tant le rapport intitulé, remis au Gouvernement le 8 octobre 2020, que la Haute Autorité de santé recommandent de mettre en place un suivi global de la grossesse, dans lequel les intervenants seraient limités et agiraient de manière coordonnée. Ce suivi est indispensable au bon déroulement de la grossesse et de l'accouchement. Je le rappelle, il est possible, pour une femme, de choisir d'être suivie, en prénatal, par une sage-femme.

il y en a, en tout cas, moins qu'avec des intervenants multiples, car la sage-femme référente tiendra à jour un dossier obstétrical complet, transmis au médecin traitant. Cela permettra, entre autres, d'aider à la construction du projet de naissance dans un climat de confiance, de faire le lien avec la maternité, d'éviter des passages aux urgences et de rendre effectif le volet anténatal du programme d'accompagnement du retour à domicile, le Prado, en organisant en amont les sorties de maternité, précoces ou non, des femmes et des nouveau-nés. Cette mesure a été élaborée en lien avec le Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Quel

Ces amendements tendent à permettre à toute assurée enceinte de déclarer à son organisme d'assurance maladie le nom d'une sage-femme référente, afin de favoriser la coordination des soins, en lien avec son médecin. La mise en place d'un professionnel de santé référent de périnatalité correspond effectivement à une proposition du rapport de la Commission des 1 000 premiers jours, remis par Boris Cyrulnik. Elle répond à un réel besoin de coordination et de suivi tout au long du parcours de natalité. Ce que nous avons prévu pour atteindre cet objectif, sur lequel,

Afin de garantir un suivi, dans la logique du parcours de soins coordonnés, un compte rendu des soins réalisés par la sage-femme sera adressé au médecin traitant et pourra être reporté dans le dossier médical partagé

d'être suivie par une sage-femme ou par un médecin généraliste ; il faut toujours revenir à cela pour bien comprendre ces amendements. Dans le cadre du suivi obstétrical ou gynécologique, la sage-femme doit

Si la patiente tarde ou ne peut pas prendre un rendez-vous chez son médecin, elle risque de subir une perte de chance ou un surcoût financier. Cette mesure a été supprimée au motif que les spécialistes vers lesquels la sage-femme pourrait orienter une patiente dans le cadre du suivi de la grossesse seraient en accès direct. C'est effectivement le cas du gynécologue,

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l'article 2 B, qui autorisait les sages-femmes à adresser leurs patientes à un médecin spécialiste sans passer par le

un rendez-vous préalable avec leur médecin traitant. Cette dérogation au parcours de soins coordonnés présentait également l'avantage de réduire le risque de renoncement aux soins,

Je partage l'avis de M. le rapporteur. Les choses ont un sens. Encore une fois, on étend considérablement le périmètre du champ d'action des sages-femmes.

veut. Le système de soins, c'est comme une maison à deux étages : on entre par le rez-de-chaussée, on monte au premier étage, puis au second ; on n'entre pas par la fenêtre du second pour sortir par celle du premier ... Il y a une cohérence

Mme Guillotin ou M. Savary. Il est vrai que, tout à l'heure, j'ai présenté un amendement tendant à ce que la sage-femme puisse prescrire des médicaments, mais, dans mon esprit, c'était en accord avec le médecin traitant. Il s'agit